j'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur est parvenu à l'adoption d'un texte commun. La parole est à monsieur Claude Raynal, président de la commission des finances, vous avez la parole monsieur le président. Bonjour, monsieur le Ministre excusez-moi je vous avez pas vu arriver un application de l'article 46 bis alinéa 2 du règlement et afin de faciliter organiser sur nos nos débats à la commission des finances demande l'examen séparé des amendements à 800 88 et 916 déposer sur la mission enseignement scolaire tout à l'heure. Merci, je suis saisie, donc en application de l'article 46 bis alinéa 2 du règlement du Sénat d'une demande de la commission des finances d'examen séparé des amendements 888 et 916 portant sur les crédits de la mission scolaire et ce qu'il y a des oppositions, je n'en vois pas, il en est ainsi décidé l'ordre du jour appelle l'examen des crédits de la mission Immigration, asile et intégration pour 2023 la parole est à monsieur Sébastien Meurant, rapporteur spécial de la commission des finances pour cinq minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, 5 minutes pour présenter un budget sur l'immigration, l'asile et intégration. Je pense que sur tous les bancs, ces sujets apparaissent comme des sujets politique majeur pour l'avenir de notre pays à l'heure des bouleversements géopolitiques multiples guerres explosion démographique, épidémie, changement climatique, nous devrions parler de frontières de souveraineté de la France et de la volonté européenne de protéger ou non les frontières extérieures de l'Union des frontières à l'extérieur pour une tranquillité publique à l'intérieur sans contrôle d'accès multiple sans caméra jusque dans nos écoles, vigiles dans tous les magasins police devant les lieux de culte pour vivre dans une société libre et apaisé au Parlement, nous devrions parler objectif chiffres Nombre savoir combien de personnes nous voulons accueillir pourquoi combien de personnes nous accueillons combien de personnes sont déboutés du droit d'Ali d'asile et combien cela coûte au pays, hélas, comme les années précédentes, ce budget n'est que le symbole de l'impuissance publique et de l'absence de volonté.

pour accueillir, soigner loger intégrer et trop doux pour ceux qui pensent que la France ne veut pas, je résume : accueillir toute la misère du monde quand on apprend cette semaine par le ministère de l'Intérieur que 93 % des vols dans les transports en Île-de-France sont le fait d'étrangers. Y a-t-il encore des personnes honnêtes pour contester le lien entre insécurité et immigration, y a-t-il encore des personnes honnêtes dans cet hémicycle. Pour contester que notre droit des étrangers est inopérant capte en plus de la moitié du droit administratif que nos procédures généreuses sont détournés par des associations militantes trop souvent financé par des deniers publics. Monsieur K stagiaire, ex-ministre de l'Intérieur, constatait la complicité des ONG avec les trafiquants, le directeur général de l'OFII écrit dans le Grand Dérangement l'immigration en face l'hospitalité national pour tous, c'est l'hospitalité pour personne, il nous faut des règles, il nous faut choisir. Depuis le début de 2022, 40000 migrants sont passés en Grande-Bretagne 30000 ont été interceptés et sauvé par nos forces de l'ordre, cela représente plus de la moitié de l'action de l'État en mer malgré tous ses efforts, des personnes se noient, prenant tous les risques pour venir dans un eldorado qu'on leur a vendu car c'est bien de cela dont il s'agit, ces personnes sont prises dans des filières criminelles organisées et nous laissons faire et subissons la loi des passeurs, ce n'est pas inéluctable, le Danemark, l'Australie, le Japon ont pris à bras le corps sans tabou ni angle mort, ces questions d'immigration de masse qui transforme et bouleverse nos sociétés les élections récentes en Suède, en Italie, les émeutes à Bruxelles où en ce moment même à Mayotte, devrait nous inciter fortement à arrêter de faire semblant, c'est notre mission de parlementaire de contrôler la politique migratoire et cela devrait être de la responsabilité du ministre de mettre en oeuvre la digue politique migratoire, or en fait de politique, nous nous voyons que la politique des petites phrases, en 2019, le président de la République déclarait vouloir exécuter 100 % des OQTF. En 2021, ce chiffre s'élevait à 6 % sur les 6 premiers mois de l'année 2022, nous sommes à 6,9 j'ai une pensée pour la petite Lola et sa famille et tout ceux qui ont été meurtries par la faillite de l'État en la matière, de Georges Marchais en 1980 qui voulait mettre fin à l'immigration illégale et au au séminaire UDF-RPR de Villepinte sur l'immigration de 1990 en passant par les innombrables déclarations ouvrages récents sur les territoires perdus de la République, l'islamisation de nos vies de la partition du territoire, nous devrions nous parlementaires nous on parie avec courage et lucidité de ces questions, mes chers collègues, l'Amicale gaulliste a reçu le 15 novembre l'ancien patron de la DGSE, Pierre Brochand son constat lucide, implacable factuel, appelle une réponse à la hauteur des enjeux qui sont immenses. Cet État qui a confiné le peuple français est incapable de savoir combien il y a d'étrangers en situation irrégulière sur le territoire, le rapport parlementaire de nos collègues gris quoi député ex-député en marche et François Cornut-Gentille, député LR nous apprenait en 2018, que l'État ne savait pas dans le seul département du quatre-vingt-treize combien il y avait de clandestins à 150000 200000 voire 400000 prêts qui avez-vous fait depuis cette réponse Monsieur le Ministre, nous ne la voyons pas dans ce budget, qui est une caricature, une de plus du en même temps je dois m'arrêter et je vous invite à voter bien entendu contre ces crédits, je vous remercie pour votre attention. Merci, cher collègue. La parole est à Madame Muriel Jourda, rapporteur pour avis de la commission des lois pour 3 minutes. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, mais mes chers collègues, l'avis de la commission des lois sur ce budget, asile, immigration, intégration a été défavorable pour des raisons diverses selon les groupes, et cela vous sera expliqué, je pense au fil de la discussion générale, c'est un budget qui comprend 2 milliards 7 ans l'autorisation d'engagement et de milliards en crédits de paiement, il est en augmentation faciale de 6 % c'est une augmentation et il a été en augmentation depuis plusieurs années, qui a pu donner un certain nombre de de solutions et apporter un certain nombre d'amélioration à la situation en France, notamment grâce à l'engagement de tous ceux qui, dans les services de l'État oeuvrent en faveur de l'accueil et en faveur de l'immigration et en tout cas de son traitement Il n'est pas suffisant d'augmenter un budget il faut examiner quel est le résultat de l'action publique suite à cette augmentation de budget sur l'immigration légale et sur l'intégration, cela correspond à 27 % du budget, nous avons des délais de traitement qui sont en augmentation notoire, il devrait être de 90 jours ils sont à 117 jours mais je dois la vérité de dire que c'est l'accueil des réfugiés ukrainiens qui a très largement accru ce délai de traitement des dossiers beaucoup trop important, nous avons 270000 délivrance de titres. De primo-délivrance, c'est-à-dire de personnes qui arrivent sur le territoire dont 31000 régularisés dans le cadre de la circulaire Valls, c'est-à-dire de personnes qui sont arrivés illégalement dans le territoire pour arriver à un stock de environ 3,5 millions de titres de personnes en situation sur le territoire, avons-nous une politique de migration légale et de migration qui ne soit pas clandestine sur ce territoire. Sur l'asile, 63 % du budget 10000 dossiers par mois 58 % seulement des demandeurs du droit d'asile qui sont hébergés des délais de traitement qui sont extrêmement importants, 336 jours alors que nous attendons devant l'Ofpra et la CNDA des délais qui devrait de 180 jours malgré l'augmentation de cent de cent ETP à l'Ofpra, qui a été connu ces dernières années et surtout 40 % d'admission définitive de personnes qui ont demandé le droit d'asile, avons-nous une politique de lutte pour ne pas dévoyer le droit d'asile et enfin l'immigration illégale 100 du budget, une situation extrêmement inquiétante, l'augmentation aux frontières de l'Europe des personnes qui arrivent dans la clandestinité, est extrêmement importante, 2021 plus 60 les premiers mois de 2022 plus 77 % pour la route des Balkans, nous sommes passés en 2 ans de 27000 personnes à 128000 personnes qui arrivent de façon illégale sur le territoire français, 124000 obligation de quitter le territoire français délivrées 7500 exécuté, nous sommes dans une situation difficile à budget c'est la traduction d'une politique l'abondement d'un budget n'est pas une politique, avons-nous une politique migratoire, légale et illégale sur ce territoire, je ne le crois pas, nous traitons les problèmes au fil de l'eau, il va falloir définir une politique, c'est ce que nous ferons, je l'espère. Merci madame la rapporteure un rappel au règlement de la présidente Assassi. merci Monsieur le Président, je fais ce rappel au règlement, suite à l'intervention de notre rapporteur Monsieur ne rend, je voudrais lui rappeler que nous sommes ici réunis ce matin pour une séance sur la mission budgétaire Immigration, asile et intégration intégration et non pour entendent une diatribe contre les musulmans contre celles et ceux qui le pensent qu'ils feront, accompagnés des migrants dans leur parcours souvent difficile de celles et ceux qui en ont une autre comment dire le sous un souci humain et humaniste et non pas un des, des, des, des éléments de langage, comme vous avez pu user monsieur meurt en en nous insultant pratiquement, nous, nous avons des responsabilités à l'égard de ces personnes, nous les assumons ces personnes et ce qui me gêne le plus Monsieur Moran, c'est que, voyez-vous, je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait le débat qui a eu lieu en commission des des finances sur cette mission budgétaire, donc j'en appelle à la raison et à la sagesse. Non, non. Oui, madame la présidente, je me permets de vous dire que c'est pas franchement un rappel au règlement, hein, non, non, madame la présidente Assassi non vous direz-vous même dans quelques minutes, que vous avez à dire, personne n'est là pour censurer les propos de qui que ce soit, que vous soyez d'accord pas d'accord, c'est une chose mais c'est pas un rappel au règlement sur l'ordonnancement de nos travaux mais. Nous en prenons acte et acte et donner de votre rappel au règlement, dans la suite non non non non de notre discussion, je vous rappelle que le temps de parole attribués à chaque groupe pour chaque unité de discussion qu'on prend le temps d'intervention général et celui d'explication de vote par ailleurs le gouvernement disposera de 10 minutes pour intervenir, la parole est d'abord à monsieur Jean-Yves Le compte pour le groupe socialiste, pour six minutes. C'est C'est le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, il est vrai que nous attendons toujours un rapport sérieux de la commission des finances sur ce budget parce que les diatribes, nous pourrons les avoir, le 13 décembre si nous estimons que c'est ça qu'il faut faire d'ici là, je souhaiterais plutôt me concentrer sur un certain nombre de 2, liés à la fois à des remarques générales et d'autre part à à l'action et au à la situation budgétaire de de de cette mission, j'espère d'ailleurs qu'avant le débat du du 13 décembre au Sénat, nous recevrons le rapport qui est prévu par la loi avant le 1er octobre de chaque année et qui rap qui qui précise les les éléments de la politique d'immigration du du gouvernement ce sera utile pour nos débats quelque 5, remarque avant de rentrer plus dans le détail sur les questions budgétaires, d'abord la France cette année, en tout cas à une demande d'asile soutenu mais beaucoup plus stable que nos partenaires européens, nous avions remarqué en 2015, nous remarquons aujourd'hui aussi face à la crise ukrainienne par rapport à ce que les eaux aux à-coups que vivent un certain nombre de nos partenaires notre schéma est beaucoup plus stable et donc bon cap en capacité d'être beaucoup plus prévisible, deuxièmement je voudrais saluer la mise en place de la protection temporaire rapidement par l'Union européenne et par l'ensemble des administrations dans les pays, les États membres de l'Union, il est important que les préfectures incite les Ukrainiens et les résidents ukrainiens vers ce dispositif plutôt que vers de la demande d'asile, et il est aussi important pour l'avenir, d'offrir une stabilité aux personnes qui sollicite cette protection temporaire dans le cas où il trouverait un emploi en France, je remarque aussi que la liberté de circulation dans l'Union et le droit de travailler immédiat que permet cette protection temporaire, produisent des effets très positifs et que ces outils doivent aussi être mis en oeuvre et réfléchi, nous faire réfléchir sur l'évolution du pacte asile migration je remarque toutefois que face aux destructions de des infrastructures vitales en Ukraine, rien n'est budgétée pour un éventuel nouvel afflux en en 2023 je, je suis de ce point de vue-là inquiétant de 3ème remarque 17000 morts en Méditerranée depuis 8 ans, c'est un drame et un échec absolu à la fois de l'Europe et de l'Afrique, un drame qui nourrit les passeurs et pour lequel une coopération et une compréhension entre les États, des 2 côtés de la Méditerranée est indispensable et je rappelle que l'action des ONG est indispensable pour sauver des vies, et que que seuls 15 % des personnes qui arrivent sur le territoire de l'Union européenne et qui débarquent sur nos plages proviennent de ces bateaux, il était indispensable de d'avoir ça en tête, enfin : la solidarité européenne, elle est primordiale, ça veut dire le respect du droit, ne pas excuser l'Italie qui refuse de respecter le droit de la mer, mais ne pas excuser la France lorsqu'elle refuse de respecter le droit de l'Union sur la délivrance des visas sur les contrôles des frontières intérieures de l'Union, oui je sais, le Conseil d'État refuse d'envoyer une question préjudicielle à la CJUE mais lorsqu'une juridiction autrichienne le fait et précise que les contrôles intérieurs dans l'espace Schengen ne sont pas conformes au droit de l'Union, la France fait comme si ne rien n'était, ce sujet est trop sérieux, Monsieur le Ministre, pour qu'entre États membres, nous fassions bac à sable, cet ensemble que nous ferons face à ces difficultés, elles sont nombreuses, que ce soit pour la Grèce pour l'Italie pour l'Espagne, qui fait face à la situation au Venezuela mais aussi pour les pays baltes et la Pologne face à la situation en Biélorussie enfreint, sur les questions d'asile il est absolument indispensable de changer de paradigme en s'inspirant de ce qui a été fait avec la protection temporaire donné va favoriser l'autonomie des demandeurs d'asile, c'est-à-dire toute de suite délivrer des cours de français et le droit au travail, c'est plus économique, et ce sont des facteurs d'intégration pour la suite, monsieur le Ministre sur ces derniers mois quelques remarques : d'abord des instructions données au poste consulaire pour les instructions de demande de VISA qui sont contraires au code Schengen VISA en particulier pour les ressortissants d'Afrique du Nord, une brasserie, une grave crise de confiance émergent entre la France et l'Afrique d'une manière générale, compte tenu de votre politique, les communautés d'affaires à l'étranger se plaignent parce que elles ne peuvent plus avoir des relations normales d'affaires entre la France et leur pays de résidence, il ne faut pas s'étonner de l'évolution de la place de la Turquie, par exemple en Afrique, si nous ne délivrons plus de visas pour des échanges normaux et de la mobilité normale entre notre territoire et les pays africains. Cette évolution vers de mobilité nouvelles, elle est à la fois une nécessité humanitaire, économique et géopolitique concernant les préfectures, il est absolument inadmissible de constater que si les files d'attente ont disparu, c'est juste de l'hypocrisie,

pour le contentieux des étrangers auprès d'ETA et plus de 55 % de l'activité des cours administratives d'appel, ce n'est pas normal, cela coûte très cher. à l'état, nous ferions mieux d'investir cet argent dans des ETP dans les préfectures pour mieux servir les demandes pour faire en sorte que les personnes qui sont en situation régulière, le reste, Monsieur le Ministre, sur les questions d'éloignement, c'est pareil, il y a un bilan à faire, ce n'est pas satisfaisant et quant aux collectivités locales, elles subissent, Monsieur le Ministre votre politique vis-à-vis des dublinés, elles doivent tous les jours. Accueillir, héberger les personnes qui n'ont pas de droits en France parce que nous n'en avons pas une politique digne vis-à-vis des dublinés c'est la raison pour laquelle, Monsieur le Ministre, compte tenu de ces éléments de critiques de votre politique, vous l'aurez compris, nous ne pouvons pas donner de moyens à une politique que nous contestons, en profondeur, c'est la raison pour laquelle nous voterons contre ces critiques. Merci, cher collègue là par les maintenant, madame la présidente Assassi. Pour le groupe CRCE pour 4 minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la mission budgétaire donc Immigration, asile et intégration pour 2023 est en hausse de 6 % par rapport au budget 2022, mais c'est encore bien loin. D'une réelle prise en compte des besoins et des enjeux en la matière, de plus, cette mission s'inscrit dans la perspective d'un prochain projet de loi gouvernemental qui sera donc présenté, si j'ai bien compris au début de l'année 2023, cela fait des années que la politique migratoire est marqué par une dégradation des conditions d'accueil et d'accompagnement par des atteintes à des droits fondamentaux, notamment à l'égard des mineurs isolés étrangers de nombreuses associations, les défenseurs des droits qui se sont succédé la Cour européenne des droits de l'homme, ainsi que des organisations internationales pointent du doigt la France pour tous ces manquements, la loi asile immigration 2018 à laquelle nous nous sommes fortement opposés n'était ni équilibrée ni efficace et elle a complexifié le droit d'asile et des étrangers, elle a ainsi accentuer la mise sous contrôle des demandeurs d'asile et multiplier les obstacles et les contrôles afin d'entraver l'accès des étrangers à leurs droits fondamentaux, les dispositifs mis en oeuvre, tels que le raccourcissement des délais de recours, le doublement de la durée de rétention n'ont pourtant pas eu l'effet dissuasif, entre guillemets, en revanche, la rétention des enfants a continué de croître les centres de rétention administrative sont saturés et l'externalisation de la politique de contrôle migratoire et renforcé s'agissant du droit d'asile, je souhaite rappeler ici que c'est un droit fondamental, profondément ancré dans notre tradition républicaine à ce type, il est tout à fait regrettable que l'une de ses institutions, l'Ofpra soit confronté depuis plusieurs années à des départs et à une forte rotation de ses agents, cette situation s'explique par la difficulté des missions confiées à ces agents par des pressions dont ils font l'objet pour accélérer l'examen des dossiers de personnes qui ont vécu le plus souvent des drames dans leur pays d'origine, la pression de la politique du chiffre, à laquelle sont soumis ces gens, ces agents influe directement sur la qualité des décisions et le recours à des cabinets de conseil privés pour réduire les délais de traitement des demandes d'asile n'a pas été d'une part des des plus appréciés par les personnels et d'autre part des plus efficaces, les personnels de la CNDA sont dans la même situation et dénonce une logique comptable dans la gestion des dossiers de la ville, par ailleurs, notons que dans la mission qui nous occupe ce matin le montant de l'allocation demandeurs d'asile a diminué d'un tiers, cette baisse est justifiée par des crédits non consommés l'an dernier, rappelons quand même que le montant de la adage s'élève aujourd'hui à 6 virgule par jour pour une personne, plus 3 quarante euros par jour par personne supplémentaires avec une majoration en cas d'absence d'hébergement, ce qui vous là, vous vous aurez demeure manifestement insuffisant pour vivre dignement, en ce qui concerne l'hébergement des demandeurs d'asile, malgré les créations de places intervenues ces dernières années, le dispositif national d'accueil pour les demandeurs d'asile demeure malgré marqué demeure marquée par un important sous- dimensionnement notre dispositif d'asile continue de souffrir d'une saturation des des dispositifs d'hébergement, il convient aussi de souligner que les autorités françaises ont le devoir d'offrir un dispositif d'accueil aux demandeurs d'asile et réfugiés et peuvent être tenus, responsable de la défaillance du dispositif national d'accueil en ce qui concerne l'état des Centres de rétention que nous connaissons bien, nous rejoignons la contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui déplore des investissements immobiliers prioritairement orientée vers un accroissement de la sécurité et non à un entretien une réfection des locaux permettant d'assurer, a minima, un accueil digne des personnes à l'occasion du futur débat sur le projet de loi pour l'asile et l'immigration, nous aurons bien évidemment l'occasion de revenir plus précisément sur ces points, mais pour l'heure, nous ne voterons pas cette mission Bureau budgétaire car elle est bien loin de répondre à des situations humaines parfois dramatiques dont les causes sont trop souvent ignorés. Merci madame la présidente de la parole est maintenant à madame. Nathalie Goulet pour le groupe Union centriste pour six minutes. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues. Je voudrais d'abord remercier notre collègue Jourda pour son rapport et et regretté que nous n'ayons pas eu monsieur le rapporteur de la commission des finances, la version de la commission des finances je rejoindrai ce qui est dit Madame Assassi tout à l'heure. Parlant de l'Ecclésiaste que vous devez connaître il y a un temps pour tout, il y a un temps pour le discours et il y a un temps pour être rapporteur de la commission des finances, donc, pour les gens qui ne sont pas à la commission des finances l'éclairage de la commission des finances nous manque, heureusement que nous avons lu le rapport donc. Monsieur le monsieur Monsieur le Ministre, j'aimerais d'abord vous interroger sur la disparition du fichier âgé de rêve qui figure. Dans les annexes de du rapport de nos rapporteur de la commission des lois, qui se sont, à juste titre, interrogé sur le projet administration numérique des étrangers en France, la disparition de ce fichier, et son remplacement par la pour un budget d'à peu près 28 millions d'euros, si j'ai bien lu m'intrigue et m'inquiète après avoir vécu Louvois et la PNIJ je suis un peu inquiète de cette disparition et j'aimerais que vous nous donniez quelques renseignements sur ce nouveau système, pouvez-vous notamment assuré que les communes, les collectivités, les organismes de Sécurité sociale on auront bien un accès à ce fichier, vous avez récemment rappelé que les personnes sous OQTF qui dépendent donc de ce fichier ne pourraient plus bénéficier de certaines prestations, il a fallu attendre une crise récente, et en même temps nous n'avons rien vu au PLFSS comment pouvez-vous aussi garantir que, avec la disparition d'âgé de rêve et le nouveau fichier à neuf il n'y aura pas de Near attribué sans vérification vous savez Monsieur le Ministre, que lorsque l'on veut dans cette maison, améliorer un logiciel ou améliorer un fichier nous tombons sous les fourches caudines de l'article 40 cas en améliorant un dispositif, nous créons une dépense même si cette dépense doit occasionner des économies il revient au gouvernement d'améliorer ses dispositifs dans la vision que nous pouvons exprimer de 9 ans dans cette maison, sur ce sujet, donc moi je suis vraiment inquiète sur ce dispositif et les et les dispositifs transitoires et j'espère que vous pourrez me donner, Monsieur le Ministre des Outre-mer quelques renseignements sur ce sujet, le 2ème point je voudrais évoquer ces Frontex parce qu'en réalité, les éléments dont on parle sont immédiatement connecté à ce qu'il se passe avec Frontex le 30 novembre le Parlement européen auditionné trois candidats pour mettre un terme à la période transitoire résultant de la démission de l'ancien directeur et donc pour mettre un terme à l'intérim de Madame Aja qu'Najah, directrice exécutive que nous avons auditionnés dans une audition commune de la commission des Affaires étrangères, la commission des Affaires européennes et de la commission des lois, le moins qu'on puisse dire, c'est que cette audition ne nous a pas rassurés, en effet, l'agence la plus puissante de l'Union européenne est sous pression depuis 2020, son ancien directeur, est accusé de complicité de violation de droits fondamentaux, il y a une enquête de l'Olaf, vous savez ça mieux que moi, donc en plus, il faut évidemment déploré les divergences existant entre les priorités de Frontex au sein des institutions européennes, comme pour le budget, ce qui a été dénoncé précédemment quelle stratégie, quelle volonté quelle priorité Monsieur le Ministre, vous le savez, le trafic d'être s'humains représentent 150 milliards de dollars, 40 millions de personnes sont touchées, dont le cinq 150 milliards oui c'est ça dont 150 me 40 millions de personnes sont touchées, donc 25 millions en situation de travail forcé, l'étude que j'ai menée dans le cadre de du livre que j'ai écrit sur le financement du terrorisme attestent que ces trafics procure entre 5 millions et 5 5 et 7 milliards de revenus par an je j'en bafouille, je suis certaine par ailleurs qu'une journée mondiale quand le temps entre le trafic d'être s'humains ne répondra pas à cette question, donc, nous sommes sur les questions de crimes transfrontaliers, il est urgent que l'agence Frontex puisse obtenir de nouveaux résultats entre janvier et septembre 2022, l'agence a enregistré une augmentation de 70 % par an des franchissements irréguliers, le nombre de franchissements illégaux, a progressé de 70 % au sein de l'Union européenne 130000 franchissement irrégulier par le corridor des Balkans autour de ces derniers mois, depuis le mois d'août 70000 franchissements illégaux ont été recensés sur la frontière, Turquie, Hongrie et Serbie, ce qui est à mettre en rapport avec le très faible nombre de retour Monsieur le Ministre, nous attendons des mesures européennes, elle conditionne en réalité un certain nombre de dispositions du droit national, or, ni l'un ni l'autre ne semble destiné ne semble décidé à avoir une stratégie volontaire sur cette question Monsieur le Ministre, qui est un irritant permanent partout dans notre pays, y compris dans des départements. Où il y a très peu d'émigration, donc c'est un sujet majeur sur lequel encore une fois, comme l'a dit notre rapporteur de la commission des lois, on a du mal à identifier une stratégie alors que c'est un problème non seulement légal mais aussi humain, ce qu'il nous faut régler et je ne crois pas que nous soyons évidemment en mesure de le faire avec ce budget, c'est pourquoi notre groupe le votera pas. Merci, cher collègue. La parole est maintenant monsieur Stéphane Ravier pour les non inscrits pour 3 minutes. Même pas une trentaine de parlementaires pour contrôler la politique migratoire du gouvernement, voilà qui est révélateur est extrêmement inquiétant, mes chers collègues, monsieur le président, Monsieur le Ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, pour bien saisir la réalité de l'action gouvernementale, il faut se pencher sur son financement, les chiffrent parlent en bien plus que les mots, la mission Immigration, asile et intégration n'est la parfaite illustration, derrière les discours, la réalité immigrationniste, et pour 2023 du ministère de l'Intérieur, la voici mes chers collègues 7 milliards d'euros pour l'immigration, soit une hausse de 34 % par rapport à l'an dernier 34 % à 1,3 milliard va à la politique de l'asile, soit 63 % du budget un quart, soit 543 millions en faveur du volet intégration 8,5 % de l'enveloppe est consacrée à la maîtrise des flux migratoires le dévoiement de l'asile qui est passé en seulement 20 ans de 38000 demandes par an, à 135000 constituent aujourd'hui une filière d'immigration clandestine de 1er plan que vous refusez de combattre, c'eût été pourtant salvateur et ô combien justifiée puisque l'agence européenne Frontex annonce pour 2022, une hausse de plus de 70 % des entrées illégales de migrants en Europe par rapport à 2021 avec 275000 entrées illégales en 10 mois seulement, du jamais vu depuis la crise migratoire de 2016, monsieur Darmanin, lui-même confessé lors de son audition par le Sénat, que 600 à 900000 clandestins étaient présents sur notre territoire, soit l'équivalent de la population de la ville de Marseille plutôt que de les alimenter, il est urgent de couper toutes les pompes aspirantes de l'immigration car selon une étude réalisée par la Africa ni au 52 pour 100 des jeunes Africains souhaitent émigrer en Europe, c'est de la survie de la France française dont il est question, désormais, mes chers collègues, vous confirmez votre Xeno, votre volonté d'accueillir toujours plus en créant des emplois à temps plein à l'Ofpra et et vous augmenter leur budget de 11 et 16 % pendant que des dizaines de milliers de Français dormiront et mourront peut être pour certains, dans la rue cet hiver que des millions de nos compatriotes ne pourront pas se chauffer, vous augmentez les et crédit pour l'hébergement des demandeurs demandeurs d'asiles de 840 millions d'euros pendant que vous réduisez la durée d'indemnisation de nos chômeurs vous augmentez les allocations des demandeurs d'asile qui Athènes est désormais 315 millions pendant que nos administrations sont à l'os vous accorder 5 3 millions à l'Ofpra, pendant que vous réduisez le pouvoir d'achat des Français chaque clandestin dans un centre de rétention nous coûte la bagatelle de 700 euros par jour le coût total des CRA dont vous voulez augmenter le nombre s'élève à 830000 euros par jour, soit 350 millions d'euros par an, la sobriété manifestement ce n'est pas pour tous de l'argent il y en a, mais pour les autres, toujours pour les autres, pas pour nos agriculteurs, pas pour les étudiants, pas pour l'hôpital, pas pour nos ports, ils sont pourtant 10 millions dans notre pays 10 millions et vous aussi, et vous vous obstinez à financer avec l'argent des Français, leurs propres disparition il est grand temps de s'occuper de nos compatriotes d'abord en présentant un budget de non, l'immigration est une loi de remigration je ne voterai pas, ce qui contribue, de toute évidence au grand remplacement du peuple de France. Merci, cher collègue, la parole est maintenant Madame Maryse Carrère pour le groupe RDSE pour 4 minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, Mesdames et messieurs les rapporteurs, chers collègues, c'est une mission dans l'examen des crédits est toujours difficile, comment savoir s'il faut se réjouir de l'augmentation des moyens accordés puisque d'un côté ceux qui migrent qui rarement leurs racines par gaieté de coeur et d'un autre notre nation rencontrent de réelles difficultés dans l'accompagnement de ces flux migratoires comme ça a déjà été indiqué les moyens de la mission augmente as un crédit de paiement qu'en autorisations d'engagement la hausse signifie-t-elle qu'une meilleure gestion se profile, où est-elle synonyme d'une dépense incontrôlable, peut-être que ces 2 idées ne s'oppose pas, toujours est-il que nous nous réjouissons évidemment de la création de nouvelles places d'hébergement d'urgence pour les demandeurs d'asile dans les centres d'accueil et d'examen des situations et dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, tout comme je me réjouis par exemple de l'augmentation des crédits de la côte de l'Action accompagnement des fois hier de des foyers de travailleurs migrants qui devrait, je l'espère être en mesure de financer l'accompagnement du plan visant à mettre fin aux habitats hors norme et indigne, il est important de permettre aux travailleurs migrants d'accéder à un logement individuel autonome et conforme aux standards actuels du logement nous tenons dans quelques arguments qui vont dans le sens d'une meilleure gestion seulement un autre sujet pose des difficultés et devrait bientôt nous occuper, je pense aux décisions d'éloignement ou d'obligation de quitter le territoire français, les OQTF voici un acronyme administratif particulièrement froid et qui semble entrer dans la dans la langue courante du débat politique, alors qu'il était encore peu connu du grand public il y a quelques temps si on ne parle jamais, des trains qui arrivent à l'heure, celui de l'exécution des OQTF s'invite hélas trop souvent dans le débat public, je dis hélas car l'invitation suis souvent un drame, mais pas seulement, on nous rapporte aussi parfois le récit de l'histoire de jeunes artisans sous la menace d'être expulsés hélas aussi parce que c'est un domaine qui est trop porteur de polémiques, de populisme d'idées reçues et de raccourcis, mais trop rarement traitée avec le sérieux, la rigueur, l'humanité, mais aussi de réalisme qu'il mérite, nous devrions bientôt nous retrouver autour de ces sujets puisque les concertations se sont engagées en vue de l'élaboration d'un projet de loi immigration nous en connaissons d'ores et déjà quelques contours possibles, le renforcement de l'effectivité de ces fameuses OQTF ou la création d'un titre de séjour métiers en tension, ce n'est pas encore le moment de parler du fond, mai sur la forme, d'autre part, le monde devra se saisir de l'occasion pour traiter ces questions dans un état d'esprit de travail de modération et de compromis, bref il faudra nourrir le débat construit et laisser de côté les invectives et les petites formules qui n'apporte rien, sauf quelques rares écarts cette dynamique que je décris et celle du Sénat, la plupart du temps, tant mieux, espérons qu'elles soient partagées au-delà de notre hémicycle, mes chers collègues dans l'atteinte de ces débats à venir, notre groupe s'abstiendra sur les crédits de cette mission, je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est maintenant monsieur Philippe Pemezec pour le groupe Les Républicains pour cinq minutes, vous avez la parole cher collègue. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Tous les ans, nous nous retrouvons sur ces bancs pour débattre des moyens donnés à l'État pour traiter de ce qui est aujourd'hui aux yeux des Français la question numéro 1, celle de l'immigration et de l'intégration des populations étrangères et tous les ans nous demande plus de moyens pour conduire cette politique, sa réflexion sur la question fondamentale : quelle politique et pour nous conduire ou. Permettez-moi simplement de reprendre les termes du ministère en 2021 dans la préparation du budget 2022. Je cite une approche adaptée et équilibrée de l'immigration, les flux migratoires reste important et leur maîtrise demeure un enjeu essentiel pour lutter contre l'immigration irrégulière avec la pluie de nos partenaires européens, la France se dote d'outils et de processus efficace en face de ses jolies promesses, nous avons mis de l'argent, beaucoup d'argent, le contribuable a mis près de 2 milliards d'euros pour quel résultat, je n'ai pas envie de tirer sur l'ambulance mais je me dois de rappeler à nos collègues de dossiers qui ont été très médiatisé sur le coup, mais dont les suites ont été beaucoup moins entendu dans les médias, d'abord le chiffre des OQTF. Suite à l'effroyable meurt de la petite Lola en octobre dernier, la question de l'exécution des obligations de quitter le territoire français a été remise sur le tapis avec un constat sans appel l'exécution des OQTF est en baisse constante depuis l'arrivée de la gauche en 2012, il était encore de 22,34 % à l'arrivée de François Hollande, ils ne sont plus que 5 virgule 67 à la fin du 1er mandat d'Emmanuel Macron, ce qui correspond à une baisse de 12 % en rythme annuel et pourtant les crédits budgétaires accordés sont là et en augmentation : plus 6 % ça été rappelé tout à l'heure pour 2023, cela prouve que ce n'est donc pas uniquement une question de moyens, j'y reviendrai 2ème sujet : l'affaire de l'Océan Viking, je n'ai pas besoin de vous raconter l'histoire, un navire de 234 migrants qui errent en Méditerranée avant d'arriver à Toulon grâce à l'humanité du gouvernement, bilan 66 personnes se sont vu accorder le droit d'asile 123 ont été interdits de territoire avant d'être remis en liberté par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la justice n'ayant pas eu la possibilité de se saisir de tous les dossiers dans les temps et concernant les 44 mineurs isolés accueillis la moitié a fui pour rejoindre leur famille dans le nord de l'Europe enfin, seules 2 personnes ont été renvoyées vers le Mali. C'est un camouflet pour le gouvernement, qui aura beau jeu de s'abriter derrière le manque de moyens de la justice et notre incapacité à faire face à la vague migratoire qui enfle, année après année, le problème est que notre système fondé sur la confiance est en train de craquer de partout, sous les yeux, consterné, des Français qui le constate tous les jours et nous reproche à nous, l'ensemble de la classe politique, cette incapacité à juguler cette vague qui envahit tout, on peut toujours discuter du nombre des cartes vitales en circulation en France le chiffre varie mais c'est entre 3 et 7 millions de cartes de plus qu'il n'y a d'habitants, on peut toujours essayer de cacher le lien entre immigration et délinquance, mais le chiffre officiel du nombre d'étrangers dans les prisons et de 24,5 % alors qu'il n'y a, officiellement, que 10 % d'étrangers en France, on peut toujours dépenser des milliards dans la politique d'intégration, mais il faut savoir et c'est le politologue Jérôme Fourquet qu'il écrit que 40 % des naissances en Seine Saint-Denis porte un prénom d'origine arabo-musulmane à ce stade, ce n'est plus une question de moyens, mais une question de volonté politique, je vous rappelle et vous avez sans doute suivi un peu l'actualité regardez ce qui s'est passé en Suède, aux dernières élections, quand la classe politique se voile les yeux sur ce qui se déroule dans son pays, ce sont les populistes qui prennent le pouvoir, rebaptisé là-bas Démocrates de Suède dans le berceau de la social-démocratie et du dans une société dite avancée, à l'inverse, au Danemark, les sociaux-démocrates ont senti le vent du boulet et ils ont fait totalement machine arrière, fermeture des frontières, lutte contre l'immigration clandestine, contrôle de l'aide sociale et du coup la confiance a été rétabli avec les dirigeants de ces formations classiques et le vote populiste a été réduit à 2 et demi pour 100 des voix, ce qui était à peu près le score de Jean-Marie Le Pen en 2 exemples à méditer, c'est donc bien une question de volonté politique et de rétablissement de la confiance, je n'ai pas le temps et ce n'est pas le lieu d'énumérer les mesures nécessaires, mais elles sont relativement simples et clairs, fermeture des frontières pour remplacer l'immigration subie par une immigration choisie, renforcement des critères d'acquisition de la nationalité, mise en place d'une véritable lutte contre la fraude sociale et le travail au noir total fermeté vis-à-vis des pays maghrébins qui nous demandent des visas et ne reprennent pas leurs délinquants fin du gouvernement des juges, en échange de véritables moyens donnés à la justice pour qu'elle puisse travailler et retrouver la confiance perdue des Français que l'on me comprenne bien mon propos n'est pas d'ostraciser toutes les personnes étrangères ou d'origine étrangère qui sont en France, bien évidemment, il y a aussi des cas individuels qui mérite que l'on fasse preuve d'humanité,

La parole est maintenant à monsieur Jean-Louis Lagourgue pour les indépendants pour 4 minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, une polémique couve depuis plusieurs années maintenant, si ce n'est plusieurs décennies, celle de la très faible exécution des obligations de quitter le territoire français, voilà 10 ans que le taux d'exécution ne dépasse pas les 20 % les 3 dernières années, il était en dessous de 7 %. Faire une loi, et ne pas la faire exécuter, c'est autoriser la chose qu'on veut défendre disait Richelieu émettre ces obligations et ne pas les exécuter, c'est affaiblir notre droit, Monsieur le Ministre, nous savons que vous faites beaucoup pour changer cet état de fait ne nous examinerons bientôt un projet de loi sur l'immigration, destiné à redéfinir notre politique en la matière, le budget consacré à la mission Immigration, asile et intégration est en augmentation, le coût de la politique française de l'immigration et de l'intégration sera en 2023 de 7 1 milliards d'euros, cette augmentation est une bonne chose car il y a fort à faire en la matière, les flux migratoires se compose de différents individus atteint cherche à améliorer la situation économique d'autres fuient les persécutions et les conflits la guerre en Ukraine a généré une augmentation des demandes d'asile à juste titre, beaucoup de nos collectivités de nos concitoyens, accueil des citoyens ukrainiens, c'est l'honneur de la France. Il apparaît nécessaire de prévoir une augmentation des moyens d'administration proportionnée à l'accroissement de ses demandes pour que nous puissions les traités efficacement et dignement, il était indispensable d'augmenter le budget consacré à la gestion de l'immigration, l'affaire de l'Océan Viking démontre que l'administration ne dépasse pas, ne dispose pas de moyens suffisants pour faire face à une telle situation, cela ne doit pas se reproduire, je veux dire que ce sujet ne concerne pas uniquement la métropole de nombreux territoires ultramarins font face à une forte progression migratoire, c'est le cas de mon île la Réunion mais aussi bien sûr à Mayotte ou encore la Guyane, l'accueil des migrants doit se faire selon un principe de solidarité, il doit être réparti bien entendu entre partenaires européens fait effectivement au niveau européen que se détermine une part importante de la politique migratoire des États. L'Union dans son ensemble est concernée par la guerre en Ukraine, elle est aussi par les flux migratoires provenant du Moyen-Orient et d'Afrique, ceux-ci avaient été fortement freinée par la pandémie, ils ont repris leur rythme à présent que la situation sanitaire s'est améliorée, l'Union européenne a pris conscience de ça, Jules Nabet vu le nerf habilité à l'égard de chantage turc, le budget de Frontex est en constante augmentation, cela ne dispense cependant pas les États membres de faire leur part l'immigration en effet un impact majeur sur la politique de nombreux pays européens : le Royaume-Uni, la Suède, l'Italie et bien sûr la France si la ville représente la majeure partie des fonds de cette mission s'éloigne, cela ne doit pas nous faire oublier l'importance cruciale de l'intégration souhaiterions que davantage de moyens soient consacrés à cet objectif, c'est en effet la cohésion de notre nation qui est en jeu, le groupe les indépendants votera en faveur de l'adoption de ce budget, qui bénéficie d'une augmentation nécessaire, il n'aura cependant fort à faire en matière d'immigration. Merci, cher collègue, la parole est maintenant à monsieur Guy Bénard Roche pour le groupe écologiste pour 4 minutes.

C'est le président, monsieur le rapporteur, c'est le ministre, chers collègues, la France ne peut pas accueillir tout le monde, si elle veut accueillir bien c'est ce que déclarait : notre président en 2019 le budget qui nous est présenté aujourd'hui pourrait faire sourire, tant il est en décalage avec ce positionnement quand on voit que les crédits octroyés pour la location des demandeurs d'asile subissent une baisse de plus d'un tiers, 36 % dans un contexte de guerre que l'on connaît, je crois, ouvrez en même temps sur la politique migratoire aussi, disait-il, toujours dans ce même entretien, augmenter l'aspect sécuritaire de la politique migratoire et en même temps, renforcer les difficultés pour des prises de rendez-vous en préfecture pour l'obtention du titre, mettre en place les défaillances du système de la CNDA manque de personnel et de moyens, et en même temps, s'appuyer sur les délais rendu trop lent pour justifier une réflexion pour modifier les règles de droit pour limiter les recours en 2017, pourtant le candidat promettait nous examinerons les demandes d'asile en mois de 6 mois recours compris c'est nécessaire pour accueillir dignement les réfugiés qui ont droit à la protection de la France, cette loi de finances illustre recule criant sur ce point, nous le constaterons lors de l'examen des Budgets des juridictions administratives pour lequel je je je suis rapporteur, vous l'aurez compris ce budget, reflet de la politique de ce gouvernement en matière d'immigration est excessivement problématique la question qui se pose désormais et qui a fait l'objet de discussions dans cet hémicycle, même lors de la présidence française de l'Union européenne et la célérité du traitement des dossiers de l'accueil permis temporaires de travailler ou logement par exemple la crise ukrainienne a montré que l'Europe et que notre pays pouvait accueillir bien accueillir et rapidement accueillir lorsque la volonté politique est mais en même temps des permis de travail pour les réfugiés ukrainiens et des arrêtés anti-repas à Calais arrêtés, jugés illégaux, il y a un mois, d'ailleurs, l'augmentation des crédits de 38 % dans le budget de cette mission pour l'augmentation des placements en centre de rétention administrative et en même temps l'enterrement définitif de la promesse d'Orléans de 2017 qui avait vu le président déclaré qu'aucun demandeur d'asile ne dormiraient dehors toujours à Calais 97 % des expulsions des lieux de vie ne sont pas suivies de mise à l'abri, c'est inacceptable, Monsieur le Ministre, je rappelle que la multiplication des crapauds répondre aux difficultés diplomatiques des éloignements est un encens non sans similaires à l'émission d'un mandat d'arrêt pour expulser une personne visée par une OQTF qui a déjà quitté le territoire 2022 le président candidat vous voulez poursuivent la refonte de l'organisation de l'asile et du droit de séjour pour décider beaucoup plus rapidement qui est éligible, et comme toujours, sous couvert de simplification ce gouvernement éloigne le demandeur d'asile du juge physiquement par exemple avec les visio- conférence et de ses droits, parfois en imposant la procédure accélérée, aller plus vite, tout le monde le souhaite mais pas au détriment des droits aller plus vite, c'est permettre, par exemple, système de rendez vous plus efficace en préfecture, je rappelle que le tribunal administratif de Paris a condamné l'OFI et la préfecture sur la mauvaise gestion de cette plateforme téléphonique pour prendre les rendez vous pour les demandeurs d'asile, on arrête, ciment de rende le numéro gratuit et de mettre en oeuvre des mesures pourraient pas plus rapidement aux appels ou sans les crédits pour cela, pour les personnels suffisants à l'écoute des demandeurs d'asile ou sans les crédits pour cela la lutte contre l'immigration irrégulière et la priorité du gouvernement, dont acte, l'action dédié a vu ses crédits augmenter de 68 entre 2017 et 2021 alors que l'action garantie du droit d'asile, pendant la même période a vu ses crédits augmenter de 12 % notre pays sonore et c'est n'orgueil d'accueillir et de sauver à juste titre, c'est l'entraîneur, je regrette que cet honneur soit variable entre l'Aquarius et l'Océan Viking, par exemple, chers collègues, n'y voyez aucune naïveté ni aucun idéalisme utopique, mais au contraire, entendez le besoin de bien accueillir, de mieux respecter les demandes des personnes arrivant sur notre sol ne serait-ce que pour leur intégration et pour l'avenir de notre pays l'acceptabilité des refus doit s'ancrer dans le respect des personnels doit s'inscrire dans le respect des procédures doit s'inscrire dans le respect des personnes qui sont accueillis une prise en charge digne de l'accueil jusqu'au traitement des demandes ce budget reflète une vision déconnectée de toutes ces préoccupations et c'est pourquoi notre groupe ne pourra pas voter, c'est crédits. Merci, cher collègue là. Par les maintenant Madame Nicole Duranton pour le groupe RDPI pour 4 minutes. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, chers collègues, il est l'heure de sortir des petites phrases politiques au sujet de ce budget Immigration, asile et intégration dont le Champ est évidemment beaucoup plus larges que les entrées illégales sur le territoire et qui par ailleurs a un budget de fonctionnement, un budget opérationnel pour traiter des phénomènes bien réels, ce n'est pas l'heure de parler de flux ou de reflux, mais bien celui de parler de personnes humaines de drames individuels devant être comme une réalité collective et avec humanité, ce n'est pas l'heure de grandes déclarations d'intentions mais celle où l'on décide de quelle façon mieux traiter l'ensemble des réalités complexes de l'immigration, en effet, cher collègue, les grands équilibres budgétaires de la mission ne sont pas déstabiliser par ce projet de loi de finances pour 2023 dont nous débattons aujourd'hui comme on pouvait s'y attendre, la commission des finances et la commission des Lois propose de rejeter les crédits de cette mission, ça a déjà été rappelé par mes collègues le montant des crédits demandés sur cette mission et sur les deux programmes qu'elle comporte, s'élève à 2. 7 milliards d'euros en autorisations d'engagement et à 2 milliards d'euros en crédits de paiement, soit une augmentation respective de plus de 34 % et de 6 % par rapport au montant accordé en 2022 près de 2 tiers de ces crédits sont fléchés vers vers la politique de l'asile, la France accueille des personnes qui vivent des drames qui sont menacés en détresse ou qui n'ont pas d'autre choix que de quitter leur pays en conflit, ce n'est pas une pratique nouvelle un peu d'histoire, elle s'inscrit dans une tradition dont les origines pourrait en surprendre plus d'un, puisqu'après la reconnaissance du principe de l'asile par Ramsès II dont le traité de Kadege en 1280 avant Jésus-Christ, c'est bien le concile des évêques catholiques réunis par Clovis à Orléans en 511 qui l'a entériné il convient par ailleurs de se réjouir de l'augmentation des moyens attribués aux 2 heures 2 opérateurs rattachés à la mission, l'Ofpra, d'une part et l'Office français de l'Immigration et de l'intégration d'autre part, avec respectivement 11 et 6 % de plus en matière d'asile, je tiens à saluer la volonté du gouvernement de redonner sa pleine porté au droit d'asile en réduisant les délais d'examen des demandes en ce qui concerne l'immigration, nous nous réjouissons d'abord collectivement de la volonté du gouvernement de rééquilibrer la part de l'immigration professionnelle par rapport à l'immigration familiale ensuite les premiers résultats positifs du dialogue avec les principaux pays d'origine, concernée par l'immigration irrégulière ouvre aussi la voie à une nouvelle Intelligence collective en la matière, enfin la poursuite de la mise en oeuvre du plan d'ouverture des places de centres de rétention administrative permettra de soulager les familles et les personnels confrontés à des situations parfois très très difficile à gérer, s'agissant de l'intégration, mes collègues et moi-même sommes satisfaits par le renforcement du vol professionnel pour le contrat d'intégration républicaine du déploiement du programme d'accompagnement global et individualisée des réfugiés, ce programme est déjà mise en oeuvre dans mon département de l'Eure, dont je me réjouis un autre motif de satisfaction et la poursuite de la rénovation des foyers de travailleurs migrants qui sont sur le territoire Eurois au nombre de 3 sur ces 3 volets, les groupes RDPI, en accord avec l'action volontaire, menée par le gouvernement, votera sans indiquer hésitation les crédits de la mission et nous sommes conscients que certains parmi vous, chers collègues, s'inscrivent dans une volonté de contribuer à l'efficacité de cette mission en affinant et retravaillant certains mécanismes financés par ces crédits, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est maintenant au dernier orateur, monsieur François Bonhomme pour le groupe Les Républicains pour cinq minutes. Vous avez la parole cher collègue. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président commission je rapporteur général, mesdames et messieurs, rapporteur, nous voici donc ce matin à l'examen des crédits de la mission Immigration, asile et intégration qui me permet d'aborder la question de l'immigration, à l'angle et sous l'angle des travaux budgétaires et avant la prochaine organisation de temps notre assemblée d'un débat à l'application de l'article 50 de la Constitution, de prime abord, je relève d'abord que les crédits de la mission connaissent une hausse bienvenue que nous voulons saluer ici en crédits de paiement comme en autorisations d'engagement ces augmentations s'inscrivent dans un contexte de forte inflation, naturellement, et plus encore de sortie désormais marquée par la parenthèse Covid durant laquelle les flux migratoires de Maurer a fortement perturbé et à certains égards, en deçà des chiffres de 2019 d'ailleurs, il convient de le relever les crédits de cette mission de tout comme tous ceux de l'Outre-mer cet après-midi d'ailleurs ne recouvre qu'une fraction, un peu moins d'un tiers des dépenses des politiques français de l'immigration et intégration et parmi ceux de la mission, la majorité un peu moins de 2 tiers est consacré à l'asile ne laissant ainsi que des portions, limitées à l'intégration et à la lutte contre l'immigration illégale dans ce contexte, la hausse des crédits de la mission n'est pas suffisante et ne saurait occulter les insuffisances des politiques traitant des questions migratoires et de l'Asie, en effet, les indicateurs souvent et malheureusement parfait dont nous disposons, révèle les difficultés croissantes que nous connaissons dans la gestion de certaines problématiques majeures, et en particulier celle de la maîtrise de l'immigration illégale, c'est ainsi que le taux d'exécution

pour 124111 prononcé, même en considérant que cet indicateur présente des faiblesses et ce que n'a pas manqué de faire le ministre Darmanin qui c'est l'engouement forcé de l'expliquer devant notre commission ce taux demeure particulièrement bas ce constat de l'existence de graves insuffisances n'est pas nouveau, nous avions relevé la chose lors des précédents Budgets, et encore récemment, la commission des lois, formuler des recommandations par le rapport de notre président, François, on a le buffet intitulé : services de l'État émigration retrouver sens et efficacité en Un tableau préoccupant du dynamisme des flux de personnes en situation irrégulière d'importantes marges de manoeuvre d'époque et de progression existe donc l'annonce d'un tableau d'un texte sur l'immigration, l'année prochaine d'ailleurs. Pas mal repoussé démontre, si besoin, si besoin est que notre nombre de chantiers demeure a lancé et que l'exécutif Anna je crois pleinement conscience, or les moyens fournis à cette mission demeure très insuffisante pour faire face aux enjeux de l'immigration de l'asile et de l'intégration, trop souvent, nous avons ici l'impression d'être dans un budget d'accompagnement de plutôt que de maîtrise des flux de l'immigration nous accompagnons de processus plutôt que le maîtriser un parallèle des interrogations par ailleurs récurrente d'un projet de loi de finances à l'autre subsistent sur la sincérité des comptes par exemple est irréaliste, monsieur ministre hein, ce contexte de de rebond post-Covid d'envisager une baisse de 36 % des dépenses de l'allocation pour demandeurs d'asile en 2023 à notre commande tout aussi plus le souligner rapporteur le traitement de la question des réfugiés irakiens s'est révélé insatisfaisant. Ceux-ci sont actuellement bénéficiaires de dispositifs de protection temporaire or malgré ce statut temporaire et les incertitudes qui entourent inévitablement la situation de guerre est né en Ukraine, l'accueil administratif et physique, l'hébergement et d'autres éléments tels que la ce scolarisation des enfants nécessite une préparation et une visibilité à maman, il paraît incompréhensible que les évaluations de la question fournit au législateur, au moment du budget soit aussi limitée, par conséquent, même si la hausse des crédits et un certain nombre d'éléments de tels que la consulter consolidation du réseau des centres de rétention admnistrative ou des locaux de rétention admnistrative. Ou l'amélioration encore des délais de traitement de de l'Ofpra, vont effectivement dans le bon sens, il n'en demeure pas moins que les faiblesses et les lacunes de la mission demeure considérable,

Je le président, mesdames, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous prie d'abord d'excuser. Le ministre de l'Intérieur des outre-mer qui ne peut être présent aujourd'hui puisqu'il est en Calédonie avec lequel ils étaient avec lui hier encore juste répondre d'un mot avant le mon discours écrit au rapporteur, personne ne peut dire que l'immigration n'est pas un sujet qui préoccupe le ministre de l'Intérieur. ça n'existe pas de dire ça, il viendra le dire en défendant la loi sur l'immigration, il vous verrez que c'est sa préoccupation quotidienne avant aussi de rentrer dans le discours, quelques chiffres pour qu'on parle de la même chose : d'un côté ou de l'autre, nombres de places autorisées pour l'hébergement des demandeurs d'asile et ces chiffres que vous avez depuis des années 82362 en 2017. 118732. En 2023. Non mais c'est pour les personnes qui sont là-bas, là, madame la sénatrice, madame la présidente, vous avez contesté ces chiffres, écoutez-les. Quant au délais de l'Ofpra. Il était de 261 jours en 2021, il est de 128 jours en 2022, d'où l'effort, nul ne peut le contester. Précisons aussi qu'il y a 26 craint CRA et 22 en métropole rentre maintenant dans le discours sur le budget Immigration Asile intégration de programme 4 pour 100 CP dans plus en 2023 par rapport à 2022 pour le porter à 2 7 milliards en à eux et 2 milliards en CP. Partant, je l'ai dit de données fiables pour éviter les fantasmes, les flux migratoires sont en progression dans le monde entier, ce n'est pas une question de France, c'est une question d'Europe, d'Amérique du monde entier. Qu'il s'agit de l'immigration, la demande d'asile dans d'autres pays compte ainsi 7 7 % de ressortissants étrangers, ce qui a donné lieu en 2021 à la délivrance de 270000 titres de séjour environ. En 2022 110615 premières demandes ont été. C'est enregistré, rejoignant ainsi des niveaux de l'année 2019 rappelons que notre pays n'a pas cessé et ne doit pas cesser d'être un pays qui respecte le droit international et qui respecte avec humanisme les situations dramatiques. De manière difficile comme on l'a vue sur l'océan de Viking puisque. Ce sont des problèmes européens nombreux. Et en augmentation, cependant, nous continuons, nous continuons à lutter contre l'immigration clandestine 170 millions d'euros prévue en 2023 soit 18 % de plus qu'en 2022. Pour mémoire, mais disons-le aussi, aucun des orateurs ne l'a dit au 31 octobre 2022 ce sont déjà près de 274 filières qui ont été 1023 passeur interpellé la politique qui se traduit dans ce budget est cohérente avec ces chiffres, avec la manière de réagir, nous continuons à mener une politique ferme face à l'immigration irrégulière, un effort sans précédent et réalisé en faveur du développement des capacités de rétention avec plus de 300000 places à l'horizon 2027 contre 1500 aujourd'hui 10 millions et plus de 125 millions d'euros prévu dans ce PLF 10 millions d'euros sont également prévues pour l'externalisation de certaines tâches non régaliennes effectuées. Sans Avantage précis par les effectifs de police frontière aujourd'hui par ailleurs dans le cas des débats sur La Lopmi, près de 60 millions d'euros seront ajoutés chaque année chaque année à la trajectoire budgétaire permettant ainsi d'augmenter les moyens dévolus à la rétention administrative s'agissant des l'éloignement des étrangers en situation irrégulière pour motif d'ordre public 3000 étrangers ont été délinquants ont été éloignés à leur sortie de détention 2021 2022 en 2 ans, plus de 2500 titres de séjour ont été retirés par les préfectures pour ces motifs d'ordre public et 7 70000 titres en fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement sur ces éloignements le ministre en parlera, ministre de l'Intérieur en parlera. Il a souhaité que la direction les étrangers en France, clarifie puisqu'on parle de sujets qui ne sont pas les mêmes, il y a les hurlements ah préoccupé à ça les départs volontaires et les départs accompagnés, il y a la France métropolitaine, il y a l'outre-mer, il est trop simple d'analyser les choses sur un seul sur. Personne ne m'en voudra, ce stade de dire un mot sur Mayotte, compte tenu de mon portefeuille ministériel la stratégie repose depuis 2019, sur le plan si Kendra qui associe une action civile et militaire 24000 étrangers en situation irrégulière ont été reconduits à la frontière l'an passé à Mayotte. 78 % de plus qu'en 2020 au 30 novembre 2022 plus de 22400 éloignements ont été réalisés Nous continuons cependant et toujours à vouloir traiter de façon objective et humaine, les demandes d'asile. Sur l'accueil et l'examen des situations plusieurs axes d'effort mérite d'être mise en avant, d'abord, les délais de traitement, je l'ai dit, ont pu être améliorée grâce à ces efforts budgétaires consentis au cours des 2 dernières années en 2020. 200 emplois supplémentaires, l'Office français à l'Ofpra ont ainsi permis de réduire le délai 170000 décision prononcée en 2020 et 2021 dans le délai d'instruction de de moi qui avait été fixé par le gouvernement, promesse tenue, alors même que les délais de recours devant la justice administrative rendent les choses plus longue et plus difficile. évidemment, le délai de traitement des demandes d'asile a un impact Direct sur le montant de l'allocation pour demandeurs d'asile, oui ça baisse d'un tiers, mais il m'écoute pas, oui ça baisse d'un tiers. Mais c'est une. à occasion obligatoire et qui en a le droit, ne l'a pas eu. Donc c'est pas la peine de dire : ah la la, on n'y arrive pas, puisqu'on y arrive, on y arrive, tout simplement, chacun de ceux qui ont droit, madame la présidente l'obtenu. S'agissant de l'hébergement 4900 places d'hébergement pour les demandeurs d'asile et 1000 places en c'est en provisoires d'hébergement pour les réfugiés vont être créées aussi le dispositif d'orientation directive régionale introduit dans la loi de 2018 permet d'orienter les vendeurs d'asile depuis l'de France qui concentre 50 % de la demande vers des hébergements en province, c'est ainsi que 16000 demandeurs ont été orientés en 2021, dans la province, première année de mise en oeuvre. Mais la politique de l'immigration est aussi le reflet d'autres types de situation : d'une part, c'est l'accueil des primo-arrivants, je pense par exemple au passeport talent au messieurs d'attractivité en faveur des étudiants étrangers, je veux rappeler à ceux qui en ont besoin que cet accueil et non seulement la marque de notre solidarité dans le développement des pays mais aussi la garantie d'un meilleur rayonnement de la France à l'étranger, c'est pourquoi, conscients de ces réalités, des moyens importants ont été attribués à la politique d'immigration dont les crédits augmentent de 24 %, je veux souligner notamment le développement progressif du programme, agir qui va globaliser l'ensemble de cet accueil, sous l'autorité des préfets de région avec des prestations donner à des associations qui ont l'habitude de faire cela, point des dédié à l'intégration des réfugiés vers l'emploi et le logement. Par ailleurs, les centres de formation linguistique proposé dans le cas du CIR sont renforcés pour améliorer la maîtrise du français, développer des formations linguistiques, maintenant nous sommes tout à fait conscients que nous avons besoin aussi en continu, en continu, parce que le monde change en continu d'adapter notre politique d'accueil d'immigration, il ne s'agit pas de pallier des manques, mais simplement d'admettre que notre monde déboule que les crises se multiplient, que nos besoins aussi se diversifie la vérité 2017 n'est pas la vérité 2022, et celle de 2025 sera encore différente parce que le monde pourra encore changer, il est donc tout à fait logique qu'au regard de ces évolutions de ses obligations nous revisitons régulièrement notre politique d'immigration et vous allez le faire dans quelques jours, c'est le projet de loi annoncé de l'aîné, 2023 par le président de la République, un mot, enfin, s'agissant du Champ international et communautaire, nous poursuivons la discussion du pacte sur l'immigration et de l'asile après les étapes franchies dans le cadre de la PFUE

Et dire au représentant du Front national que le grand remplacement d'âge et de rêve par la nef est effectivement en place en 2023 voilà, mesdames, messieurs les sénateurs, je pense que le budget que nous vous proposons et juste. Au regard de cet équilibre très complexe entre le respect de nos valeurs républicaines, avec lequel nous ne pouvons pas transiger avec nos impératifs de sûreté qui sont notre obligation vis à vis de nos concitoyens mais aussi nos impératifs de solidarité à l'égard de pays amis à l'égard du rayonnement que nous cherchons à voir et à répondre aussi aux besoins de nos sociétés en matière de main-d'oeuvre, c'est un équilibre le gouvernement pense qu'il est atteint à ce stade, dans le projet que vous avez décidé de ne pas voter malheureusement. Merci, monsieur le Ministre, malheureusement c'est le Parlement qui en décident. Et pas. Et pas. Cas pour le moment la République étant ce qu'elle ait laissé le Parlement libre de faire ce qu'il veut, merci monsieur le Ministre. Je vous rappelle que pour cette mission, la conférence des présidents a fixé la durée maximale de la discussion à une en conséquence, si nous n'avions pas terminé l'examen de cette mission à 12 heures 30, celui-ci se poursuivrait à la fin d'émission de cette semaine et nous passerions à l'examen de la mission, pouvoirs publics. Nous attaquons immédiatement le débat sur les amendements, en commençant par le 826 monsieur Bena Roche. alors qu'une estimation établie à 135000 les demandes d'asile pour 2023, le budget de l'allocation pour demandeurs d'asile, baisse de 176 millions d'euros en 2023 amputé 36 pour pourrait être 314 millions d'euros pour expliquer cette chute, le ministère de l'Intérieur, explique que les délais d'instruction sera simplifiée pour faire des économies, avec un renforcement de la lutte contre les fraudes, donc en fonction de résultats hypothétiques et le budget est baissé par anticipation le bleu budgétaire ne fait même pas mention des réfugiés ukrainiens qui bénéficient de cette même allocation cette baisse drastique est un choix purement politique, Monsieur le Ministre, qui traduit la marque des orientations sécuritaires voulue par le gouvernement, au détriment de l'accès au droit et à la solidarité, une baisse qui est difficilement justifiable au regard des conflits internationaux et de la guerre en Ukraine le problème engendré par la sous-budgétisation de l'ADA ne fera qu'accroître les difficultés quotidiennes de personnes en détresse et que la France a l'obligation d'accueillir et de traiter avec dignité, contraint par les règles de recevabilité financière prévue à l'article 40 de la Constitution et pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, les auteurs de cet amendement à bord de l'action, garantie de l'exercice du droit d'asile du programme 303 immigration et asile à hauteur de 80 millions d'euros et baisse du même montant, l'action 11 accueil des étrangers primo-arrivants du programme 104 intégration et accès à la nationalité française. Merci, avis de la commission, monsieur La commission demande un retrait ou sinon avis défavorable et sur l'ensemble des amendements, par cohérence puisque la Commission a demandé de rejeter l'ensemble de des amendements

et donc la loi arrive bien nous verrons la loi pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose comme acte là je suis d'accord avec mon collègue mais la roche sur l'optimisme du du gouvernement mais cet optimisme semble effectivement très, trop optimiste donc, malgré tout, comme je vous disais moi nous souhaitons le retrait ou le fait que cet amendement soit soit

et que nul ne dit que celui qui a droit, ne l'a pas eu et ce sera demain comme hier, donc, si le gouvernement estime les services estime que c'est suffisant compte tenu du délai, la réduction des délais que cette prestation obligatoire, elle sera servie où le budget sera modifié ultérieurement.

Cet amendement vise à créer un fonds destiné à l'accompagnement et au suivi psychologique et psychiatrique des personnes exilées arrivant sur le territoire français, la santé mentale et plus particulièrement la souffrance psychique est un angle mort des politiques publiques concernant les personnes exilées lors de la prise en charge des primo-arrivants, les professionnels constatent que les personnes exilées sont atteints de troubles psychiques multiple en effet de nombreuses personnes subissent de leur situation pré-migratoire à leur arrivée, de multiples situations traumatisantes, les violences ayant causé leur départ, les ruptures souvent brutales que cela occasionne et le parcours d'exil lui-même semé de violences et de pertes cause des troupes si grave, renforcée par la grande précarité sociale et administrative vécu à l'arrivée, la forme la plus courante de ses troupes les le 7 Rome psycho-traumatique cette infection complique les témoignages devant l'Ofpra et le CNDA qui nous le signale notamment en raison des troupes de la concentration et de la mémoire qui affectent la capacité des demandeurs d'asile à mettre en récit leur parcours d'exil, ces derniers peuvent oublier jusqu'au prénom de leurs enfants, le stress des entretiens décuple généralement ces effets désemparés face à ce phénomène, plusieurs organismes ont signalé la multiplication des cas de suicide et demande la création de suivi psychosomatiques de ces personnes dès leur première mise en relation avec les centres d'accompagnement, c'est donc le sens de notre amendement le fort que nous proposons de créer financerait l'emploi des professionnels de santé étant psychologue, psychiatre spécialisé dans la prise en charge des pathologies traumatiques au sein des centres et géré par l'État et des organes associatif habilité à prendre en charge les personnes exilées le financement de cette mesure se ferait par transfert de 10 millions d'euros depuis l'action 03 attitude lutte contre l'immigration irrégulière du programme 303 intitulé Immigration et asile vers faute de soutien à l'accompagnement

de cet amendement et de la nécessité certainement d'accompagner d'immigrants qui viennent pour certains de zone de guerre et qui ont vécu effectivement des causes des situations extrêmement douloureuse, voire tragique et on peut se poser la question de de la dangerosité de laisser des personnes qui arrivent venant d'Afghanistan ou d'ailleurs et et je pense que les les attaques, il est l'insécurité, les attaques au couteau que nous voyons multiplié depuis ces 30 dernières années sont évidemment liés à cela et peut-être une insuffisance de moyens, mais nul ne conteste aussi que le gouvernement d'une manière générale augmente les moyens, vous l'avez vu les chiffres augmentent, mais ils ne sont pas à la hauteur des besoins qui sont immenses, la seule question qui se pose vraiment, c'est qu'est-ce que vous non, nous en avons les moyens en France, dans mon département, il se trouve que il y a un hôpital psychiatrique, le seul qui est condamnée à la fermeture et la filière psychiatrie psychologie en France est une filière qui manque cruellement de praticiens et d'étudiants, malgré tout, vous avez compris que moi je me plante dans les réalités et que je vous appelle effectivement à voter contre cette bonne intention, mais que je ne vois pas concrètement ce pouvoir se faire merci avait du gouvernement, monsieur le ministre. L'ancien préfet que je suis aurait pu aimer cette administration administrante et s'occupant de tout, et réalité, c'est que quel que soit le sujet, l'acuité rapporteur l'a dit, hein, de ce sujet compliqué de le faire faire par l'administration et par un fonds spécialisé mais pour réconforter ceux qui souhaitent cette action comme je la souhaite, je précise que ce sont environ 3 millions et demi d'euros de subventions qui sont donnés à des associations qui s'en occupe le sujet me paraît donc financer et le gouvernement émet un avis défavorable. Merci, je vais mettre aux voix le 827 avec 2 avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Aurore. Merci, c'est, c'est c'est agréable de constater que tous ces amendements font preuve de bonnes intentions qu'il faudrait appliquer mais qu'en fait on n'en a pas les moyens, donc en fait à un moment donné, si on en a pas les moyens, Monsieur le Ministre, vous, monsieur le rapporteur, si effectivement que l'autre politique migratoire et hors sol totalement, il faudrait peut-être tirer cette conséquence bon sur l'amendement 825 cet amendement du groupe écologiste solidarité territoires a pour objet d'augmenter le budget dédié à l'hébergement d'urgence pour les demandeurs d'asile, ce qu'on appelle H. selon l'avis des rapporteurs madame Muriel Jourda et monsieur Philippe Bonnecarrère sur la mission Immigration, asile et intégration le développement capacitaire du parc d'hébergement du dispositif national d'accueil a connu un coup d'arrêt en 2022, alors que là LFI pour 2022 prévoyait la mobilisation d'une provision exceptionnelle de 20 millions initialement destiné à couvrir un éventuel dépassement de la DA pour financer 4900 places d'hébergement supplémentaires ces crédits supplémentaires ont finalement été utilisés pour financer l'accueil des déplacés ukrainiens, les créations de places ont été reporté à 2023 conférence de faits à caractère d'année blanche à 2022 en 2023, de nombreux demandeurs d'asile continueront donc, faute de places disponibles dans les JDA de solliciter un hébergement en dehors des structures d'accueil et notamment au sein de structures de structures d'hébergement d'urgence de droit commun. Qui sont elles-mêmes, bien entendu, vous allez me répondre : on n'a pas les moyens puisqu'elles sont elles-mêmes pleines l'hébergement de type H UDA et pourtant capital puisque certaines places d'H. UDA sont notamment spécialisé pour prendre en charge des femmes victimes de violences ou de la traite des être s'humains, de ce fait, il nous paraît primordial de créditer davantage ses Budgets, en augmentant la part qui revient à ce type d'hébergement. L'amendement visant à transférer 5 millions d'euros d'un E et de CP de l'action 03, lutte contre l'immigration irrégulière du programme 303 immigration et asile pour aborder la création d'un nouveau programme appelé moyens supplémentaires pour l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile.

La question c'est que toujours elle, elle était toujours le même, nous traitons les conséquences et pas les causes qui est le nombre de personnes à loger et il suffit d'ouvrir les yeux à Paris et ailleurs pour voir des personnes provenant certainement de l'étranger, qui n'ont pas de place en logement et différentes sortes Huda Cada et autres et qui se trouve à la rue ou l'élu local que je suis dans des places d'hôtel puisque les départements sont amenés à et réserver des places de des chambres d'hôtel la question, c'est que nous avons pour ce budget 2023 emprunté 270 milliards d'euros que nous allons le par franchir les 3000 milliards de dettes le pouvons-nous, je vous dis non, donc je je vous appelle à voter contre cet amendement, qui est plein de bonne volonté, encore une fois, mais la politique ce n'est pas la bonne volonté, c'est des faits et on n'est pas dans les l'idéologie merci. Merci à vie du gouvernement Monsieur le Ministre. Rappeler aux sénateurs que ce budget pour l'hébergement et de 395 millions d'euros, donc là, vous proposez de rajouter 1 virgule 25 %, c'est un geste demande politique et avec ses 395 millions le PLF 2023 prévoit 4900 places nouvelles dans les DNA, un mot pour répondre au rapporteur de la commission des finances sur des UDA il y a bien les CES, les UDA il les

et d'en garder UDA pour des sujets spécifiques, un certain nombre de personnes en asile, un certain nombre de de de femmes isolées de personnes dans des difficultés particulières donc à côté de cette augmentation du nombre global de place dans le DNA, il faut souligner, je le fais avec plaisir cette clarification entre laisser à ES les H UDA et les Cada, c'est absolument nécessaire quant à l'effort, il est fait. Merci, hé bien. Qu'est-ce qui se passe c'est c'est les sigles qui vous met dans cet état, oui je m'en doutais mais Monsieur le Ministre, c'est très bien, la réponse est plus courte, allez.

Rejeté 2 amendements identiques : le 828 Monsieur Bénard Roche. Merci monsieur le président, monsieur le rapporteur, la politique, c'est la volonté politique aussi, donc, si, si la volonté n'est pas politique, je ne sais pas ce qu'est la politique, en fait, deuxièmement, Monsieur le Ministre, gouverner, c'est à peu prévoir quelque part donc en fait quand on est obligé de dépenser beaucoup plus d'argent, parce qu'on n'a pas prévu un certain nombre de choses, en fait, c'est pas des économies, excusez-moi de le dire : ça nous coûte beaucoup plus cher au final, les politiques actuelles nous coûte beaucoup plus cher que si on prévoyait un certain nombre de choses dont celles dont j'ai parlé, il faut que j'ai fait ces remarques dernière amendements que je défendrai le c'est un amendement qui vise à ouvrir les cours de français aux personnes étrangères exclu du parcours d'intégration du contrat d'intégration républicain, le fameux CIR, vous connaissez ce ce contrat d'intégration républicaine qui est conclu entre l'État français tout trop gênant en Europe admis au séjour en France avec un parcours personnalisé d'intégration concernant une formation linguistique, nous ce que nous demandons, c'est qu'un certain nombre de personnes étrangères qui existent, elles sont là, hein, c'est pas, c'est pas pour les créer, ça va pas faire un appel, une création du je ne sais pas quoi qui ne sont pas signataires du CIR et qui ont des besoins et on leur demande et à juste titre d'apprentissage de la langue française, ne serait-ce que pour sa série en France pour renforcer pour pour éviter leur précarité sociale pour éviter leur donne accès à un certain nombre de droits en demande donc à titre d'expérimentation, une ouverture de l'accès à la formation, l'acoustique pour ce public étranger, qui n'est pas signataire du CIR amendement sur sur sur sur sur l'augmentation de 200000 euros de l'action 12 au sein du programme intégration et accès de la nationalité française et une baisse de 200 équivalent de l'action 03 du programme Immigration et asile merci madame la présidente, a seize. Très rapidement, monsieur le président, parce qu'il a été très bien défendu près près précédemment, je voulais simplement redire ici que pour mon groupe, nous avons toujours souligné que la connaissance de la langue française et et l'une des conditions d'intégration en France, qui est d'ailleurs exigé par l'administration et donc cette exigence va se retrouver au coeur du projet de loi que j'évoquais tout à l'heure dans mon, dans la discussion générale donc, projet de loi immigration qui devrait être présenté en début d'année 2023 et donc sans moyens mis en oeuvre pour l'apprentissage de la langue, cette exigence peut devenir discriminatoire, voire pire encore un prétexte d'un d'un d'invisibilisation, des étrangers, voire d'exclusion, donc je pense qu'il est important de voter cet amendement alors que nous débattons justement du budget pour l'année 2023 années où nous allons débattre de ce futur projet de loi. Merci à vide de la commission sur ces deux amendements identiques. Alors déjà c'est, c'est une bonne chose de se dire entre nous que par les le français, une des conditions de l'intégration parfois on on pourrait en douter, donc c'est une excellente chose par contre 200000 euros, vous comprendrez que, évidemment, c'est plus ce également de de relève du domaine de la bonne intention et je voudrais dire à la présidente Assassi que je l'invite à écouter ce que j'ai dit tout à l'heure, il n'y avait rien de d'insultant, il n'y avait rien d'ostracisant je l'ai connu beaucoup moins idéologue lorsque la commission d'enquête sur McKinsey et moi ce qui m'intéresse, ce ne sont simplement que les faits, lorsque je parlais tout à l'heure de la, de l'insécurité et des Liens avec l'immigration, et tout le monde le dit le président le dit le ministre de l'Intérieur, le dit : il suffit de consulter tout ce qui relève des faits et pas de l'idéologie, alors c'est peut-être d'avoir évoqué, paix à son âme, Georges Marchais,

Sur ces deux amendements, je rappelle que tous les étrangers en situation régulière et qui souhaitent s'installer durablement bénéficie, vous l'avez rappelé du cours de langue dans le cadre du contrat d'intégration républicaine, le bien nommé, par contre pour les autres, je suis tenté soit de dire que c'était en dehors de la loi, soit que c'est déjà fait un certain nombre d'associations financées par l'État s'occupe activement de toutes ces personnes et des cours de français, pourquoi essayer de faire des choses qui sont déjà fait et de le faire de manière contestée, donc le gouvernement donne un avis défavorable. Merci, je vais donc mettre aux voix, ces 2 amendements identiques avec 2 avis défavorables qui est pour. Merci qui est contre. Qui s'abstient. Ils sont rejetés, enfin le 922 madame la présidente. qu'on fasse l'amalgame entre les migrants et la délinquance, on aura l'occasion d'y revenir, mais je trouve que ses propos sont inadmissible, inadmissible. Voilà, j'en viens à mon amendement, oui, oui, ben, on aura l'occasion d'en reparler avec cet amendement, nous. Souhaitons relayé une revendication qui ne va pas plaire, mais qui est porté depuis une quinzaine d'années par les luttes des travailleurs été travailleuses sans papiers que dont beaucoup sont exploités, celles-ci ont mis en lumière un véritable système qui poussent à la clandestinité depuis l'Automne 2021 3 grèves de travailleurs sans-papiers se sont successivement déclenché il dit. Tous ces toutes les conditions infernales dans lesquelles les employeurs, les fonds ou les les ont fait travailler pour certains d'entre eux, y compris pendant la Covid décidé de les régulariser, ce n'est pas fermé les yeux sur ce système, bien évidemment, qui, dans la clandestinité s'arrange une armée de réserve, c'est aussi reconnaître leur rapport dans notre société, comme sur le marché du travail, c'est enfin une mise en garde à ses patrons qui s'accommode trop facilement de cette situation.

Et vous souhaitez régulariser les sans-papiers. C'est assez étonnant venant de ce parti de l'hémicycle, de se retrouver sur la même ligne que le je parle avec des mots, vous comprendrez avec le grand capital.

je suis défavorable et et je me permettrais quand même quelque chose, monsieur le président, parler de Mayotte, ce le ministre Mayotte, la population de Mayotte, puis la moitié de la population plus ou moins clandestine. Et la moitié de cette moitié et récemment arrivé sur sur l'île et pose d'infinis problèmes en matière de sécurité en matière de travail et là on cherche effectivement beaucoup de travail pour les Mahorais et et ça pose évidemment un certain nombre de problèmes à Mayotte dans d'autres départements, également, j'ai pas cité la Guyane et pour le département que je connais bien et certain nombre de collègues ici le procureur général à la rentrée de septembre, parlait de sensibilisation du département et c'était pas un signe positif dans sa bouche, bon vote contre. Monsieur le président, puisqu'il s'agit que d'un amendement d'appel comme on dit, pour respecter le Parlement, à respecter le travail du gouvernement sur ce texte, je pense qu'il faut s'en remettre à la loi immigration qui va arriver en décembre j'mais donc un avis défavorable à ce stade. stade. Et Pepette allez, chacun s'exprime calmement Monsieur le comte. Oui, merci Monsieur le président, Monsieur le Ministre, il serait peut-être pas inutile malgré tout de ne pas attendre la prochaine loi pour que les préfectures puisse toute recevoir les demandes de régularisation exceptionnelle au séjour qui parfois ne peuvent plus être déposées, compte tenu de la situation des préfectures, déjà, ça serait un point positif, et, deuxièmement, je rappellerai que toute régularisation permet à une personne qui travaille qui cotise mais qui n'a pas les droits qui sont engendrés par ces cotisations de revenir dans une situation de droit commun et que la régularisation et le meilleur moyen d'éviter le dumping des salaires, la régularisation, c'est ce qui permet d'assurer l'égalité et aussi la croissance économique est quand même indispensable à notre pays. Merci, allez.

J'ajouterai à ce qu'a dit mon collègue monsieur le comte que en cette période de tensions dans certaines professions, il serait très adéquat de de régulariser un peu plus

de rejet des migrants et à un moment où on en a tant besoin pour certaines professions, comme je l'ai déjà dit merci. Qui est contre. Qui s'abstient. Il est rejeté, je vais procéder au vote des crédits de la mission Immigration, asile et intégration figurant à l'état B je n'ai été saisi d'aucune demande d'explication de vote avant l'expiration du délai limite je vous rappelle que la commission des finances, est défavorable à l'adoption des crédits de cette mission, qui est pour. Merci qui est contre. Merci, ils sont rejetés, merci monsieur le ministre.

l'ordre du jour ah. Appel l'examen des crédits de la mission, pouvoirs publics, de la mission Conseil et contrôle de l'état de la mission Direction de l'action du gouvernement et du budget annexe Publications officielles et information administrative du projet de loi de finances pour 2023. Vu le temps, je pense qu'on va faire passer tous les rapporteurs, on verra si on peut rentrer dans la DG après ça m'étonnerait. La parole est d'abord à monsieur Jean Michel Arnaud, rapporteur spécial de la commission des finances pour cinq. vous avez la parole un collègue. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, comme vous le savez la loi organique relative aux lois de finances prévoit qu'une mission spécifique regroupe les crédits alloués sous forme de dotation aux pouvoirs publics pour lequel le juge constitutionnel, a rappelé le principe d'autonomie financière qui relèvent de la séparation des pouvoirs. Les institutions relevant de la mission, pouvoirs publics, confrontés à des exigences croissantes d'efficacité d'exemplarité, participent à l'effort de redressement des comptes publics puisque, depuis plus de 10 ans, la dotation a progressé d'un montant nettement inférieur à celui de l'inflation constatée sur la même période pour autant en 2023, il est prévu d'augmenter cette dotation, bien que de manière modérée ainsi dans le contexte inflationniste que nous connaissons et en raison de la volonté des différentes institutions de préserver un niveau élevé d'investissement, le montant des dotations consacrées aux pouvoirs publics est en augmentation de 2 76 % par rapport à 2022, pour s'établir à un peu plus de un milliard d'euros. Commençons par la présidence de la République, après 3 années de stabilité, la dotation affectée à la présidence de la République augmente de 4 9 % c'est le vent un peu plus de 110 millions d'euros. Je signalerai parmi les faits notables, les dépenses de la présidence de la République font face, notamment après un ralentissement de la de la, de l'activité liée à la Covid 19 à une reprise des missions internationales et comme nous le verrons pour les autres institutions, des dépenses de fonctionnement, soumise à une forte inflation, malgré cela, la présidence de la République souhaite maintenir ses investissements comme ça nous a été rappelée lors de nos éditions, notamment auprès du directeur de cabinet du président de la République, Patrice, il s'agit notamment en matière de sécurité informatique ou d'économie d'énergie, un effort particulier est porté par la présidence de la République, je pense en particulier au projet de géothermie qui est en cours de déploiement dans les jardins de l'Élysée pour celles et ceux qui les fréquente assidûment jeter un oeil, d'un montant de 1 virgule 4 millions d'euros, il devrait ainsi réduire les émissions de 80 pour 100 de CO2 pour la seule présidence de la République et les pas Élysée concerne à présent les dotations des assemblées parlementaires, la hausse octroyer cette année représentent 3 35 % pour l'Assemblée nationale, et de 28 % pour le Sénat des dotations s'élève ainsi respectivement à 571 millions d'euros, donc pour l'Assemblée nationale et 346 millions d'euros pour le Sénat, j'évoquerai ici dans cette belle maison principalement notre budget, celui du Sénat, dont les dépenses augmentent de 1 virgule 18 % les charges de fonctionnement augmentent quant à elle, de 6 % en raison pour les 2 tiers de l'inflation et pour un tiers du renouvellement sénatorial de 2023, tandis que l'effort d'investissement après une année où il a été exceptionnellement élevé 33 millions d'euros, celui-ci, ramené à 17 25 millions d'euros, soit une baisse de 48 % il servira notamment à des projets d'envergure tels que la restauration des façades et couverture des pavillons Est-du palais concernant les chaînes parlementaires leur budget augmente légèrement d'un peu moins de 1 % à 0 virgule 6 % celui de LCP Assemblée nationale connaît une hausse de 1,2 pour 100, le budget de Public Sénat étant reconduit à l'identique, terminons par le Conseil constitutionnel et la Cour de justice de la République, le Conseil constitutionnel, voit certes son enveloppe se réduire de 16 virgule 71 %, pour s'établir à 13,3 millions d'euros, mais cela fait suite à une forte augmentation l'année dernière en raison des élections présidentielles, parmi ces dépenses, les moyens consacrés au contrôle des normes représentent 62 % de la dotation et sont en augmentation par rapport à l'année dernière, ceux qui sont cohérents, au moment où se déploie le portail de référence de la question prioritaire de constitutionnalité concernant, pour finir, la Cour de justice de la République sa dotation est identique à celle de l'an passé à hauteur de 984000 euros, l'été 21 avait été notamment marquée par un nombre de plaintes sans précédent qui avait dépassé lié évidemment à la situation Covid et notamment des opérations groupées, menée par certains cabinets d'avocats qui avait donc dépassé plus de 20000 plaintes depuis 2022, le phénomène s'est nettement ralentie, le nombre de plaintes s'élève en effet à 349 depuis le 1er janvier 2022 au vu de l'ensemble des éléments que je viens de vous présenter, je vous propose, avec évidemment l'avis favorable de la commission des finances d'adopter les crédits de la mission, pouvoirs publics, je vous en remercie. Merci, cher collègue, la parole est maintenant avec Monsieur Christian. Rapporteur spécial de la commission des finances pour cinq minutes.

Monsieur le président, monsieur le ministre. Je suis rapporteure chers collègues en masse budgétaire la mission Conseil et contrôle de l'État est une petite mission puis je connais crédits demandés pour 2023 s'élève à 800 du 7 millions d'euros là ne demeure pas moins une importance fondamentale pour notre État de droit, dès lors que les composés essentiellement des crédits des juridictions administratives et financières, l'efficacité de contrôle des actes de la plus à public dépendante de la d'autres actions de cette mission, celle-ci doit être suffisante et adaptée aux enjeux contemporains, notamment au volume contentieux qui ne tarissent pas, loin s'en faut, ainsi, il apparaît que la mission est intrinsèque commun liés à l'exercice des fonds de quand régaliennes de l'État. Le budget du Conseil économique, social et environnemental relève également de cette mission, mais ils ne représente que 5 % des crédits pour l'année 2023 Angola peut dédiée leur participation aux citoyennes et de 4,2 millions d'euros, notamment pour l'organisation de la Convention citoyenne sur la fin de vie, je tiens à saluer ici thermos l'internat ondulation des procédures de par jour citoyenne qui devrait permettre de diviser les coûts de par de cela illustre une nouvelle fois l'efficacité de l'État à moindre août par rapport au recours aux cabinets de conseil, comme l'avait été, j'aime mis en lumière les travaux de la commission d'enquête de chaleur si les crédits en hausse de 8 vers le 5 % par rapport à l'an passé, corrigé de l'inflation, simplement ce n'est en réalité que de 4 % soit du même ordre que la loi de finances,

par ailleurs, le volume de la mission est largement titulaire des moindres variations qui peuvent affecter les dépenses de personnel qui représentent 80 % des crédits demandés

En est-il, il faut ajouter une revalorisation vont indemnitaire à des magistrats administratifs et financiers, qui a été décidé pour maintenir l'attractivité financière de ces corps par rapport au nouveau corps des administrateurs de l'État issu de la réforme de la haute fonction publique l'alignement d'un traitement et d'autant plus nécessaire que l'obligation de mobilité a été accrue pour les magistrats administratifs concrètement la revalorisation qui vaut environ 8000 euros annuels pour les magistrats de 1er grade et 6000 euros annuels pour ceux du 2ème grade, un mot sur la mobilité de la haute fonction publique, la mobilité au sein du ministère, c'est la mobilité d'une rue à l'autre du 7ème arrondissement, la mobilité des magistrats, c'est changer de région, avec tout ce que ça implique pour la vie familiale, le travail du colon et cetera, donc ça mérite la refouillé la mobilité n'est pas la même dans toutes les administrations de l'État, vous le voyez bien, mes chers collègues, derrière la hausse des crédits de la mission Conseil et contrôle de l'État faut cachent des hommes et des femmes, et essentiellement des magistrats administratifs et financiers qui pourront exercer au mieux les missions de service public autre confié je leur raison pour laquelle mes chers collègues tout le bénéfice de ces observations, la commission des finances ou propose d'adopter les crédits de cette mission, le vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est maintenant Monsieur Paul Toussaint Parigi, rapporteur spécial de la commission des finances pour cinq minutes. Monsieur le président, Monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs pour avis, mes chers collègues, la mission Direction de l'action du gouvernement de telle qu'elle nous est présentée cette année connaît un rétrécissement attendu de son périmètre puisque l'un de ces 3 programmes a été supprimé, il s'agit du programme relatif à la présidence française de l'Union européenne qui s'est achevée le 30 juin 2022. Corrigé de cette importance importantes mesures de périmètre et de l'inflation, la mission voit ses crédits augmenter de 3,5 % en crédits de paiement et 9 % en autorisations d'engagement, il s'agit d'une hausse non négligeable qui doit néanmoins être relativisé puisqu'elle ne représente en valeur absolue et hors inflation que 30 millions d'euros en crédits de paiement et 73 millions d'euros en autorisations d'engagement ces nouvelles dépenses semble en outre justifié puisqu'elle reflète la priorité accordée par le gouvernement à la cybersécurité et dans une moindre mesure à l'écologie 2 enjeux dont l'actualité ne cesse de nous rappeler l'importance, le nombre de cyber attaques touchant aussi bien l'État que les collectivités territoriales, des entreprises ou encore bien des hôpitaux, on a vu récemment à l'hôpital de Corbeil-Essonnes, a en effet triplé en seulement 2 ans, dans ce contexte, les renforcements de moyens alloués à la cybersécurité apparaît nécessaire afin de mieux prévenir ces attaques et d'aider les organismes touchés à y faire face, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information bénéficiera ainsi en 2023 d'un schéma d'emplois 2 46 ETP supplémentaires ainsi que d'une nouvelle dotation de 25 millions d'euros afin de lui permettre d'acquérir de nouveaux locaux à Rennes. L'écologie apparaît ensuite comme un second temps je justifiant la hausse des crédits alloués à la mission Direction de l'action du gouvernement avec la création du secrétariat général à la planification écologique dont les moyens sont définies par le présent projet de loi ce nouveau secrétariat et placée directement sous l'autorité de la Première ministre, ce qui témoigne de la prise de conscience de la nécessité d'inscrire l'écologie comme une priorité transversale de l'action publique, il aura pour mission d'assurer la coordination interministérielle de l'ensemble des politiques publiques visant à assurer la transition écologique du pays et il disposera pour se faire de l'appui d'une équipe de 15 ETP TP et d'un budget de fonctionnement de 500000 euros en 2023, cela peut sembler peu au regard de d'immensité de la tâche que représente la planification écologique d'un pays de 68 millions d'habitants, mais nous attendons de ce secrétariat qu'il monte en puissance ces prochaines années afin de tenir la promesse de faire de la France une grande nation écologique je terminerai mon propos par quelques mots sur le budget annexe Publications officielles et information administrative ce budget annexe tire principalement ses ressources des recettes d'annonces légales qui dépendent fortement de l'activité économique pour cette région, le projet de loi des finances de 2023 prévoit une hypothèse de de recettes prudente à la hauteur de 167 millions d'euros, soit une baisse de 7 millions d'euros par rapport aux recettes estimées pour l'année 2022, malgré cette prévision prudente le budget annexe devrait dégager en 2 vingt-trois un nouvel excédent, estimé à 14 millions d'euros grâce notamment à la maîtrise renouvelée de ses dépenses de personnel à la lumière de ces différentes observations laquelle la commission vous propose donc d'adopter les crédits de la mission Direction de l'action du gouvernement ainsi que les crédits du budget annexe Publications officielles et information administrative, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est maintenant monsieur Olivier Cadic, rapporteur pour avis de la commission des Affaires étrangères pour trois minutes. Monsieur le président, chers collègues, la vie sur les crédits du programme 129 que nous allons vous présenter avec mon collègue Mickael Vallet porte sur la coordination de la sécurité de la Défense et plus précisément sur la cyberdéfense et les stratégies d'influence que le président de la République vient d'élever au rang de nouvelles fonctions stratégiques lors de son récent discours à Toulon, l'enjeu de la guerre informationnelle que j'avais mentionné lors des débats sur la LPM en 2018 et enfin pleinement reconnue et je m'en félicite, j'avais salué la création de Viginum l'an dernier, mais je reste circonspect en observant le Champ restreint de ses missions, qui s'arrête à la caractérisation de situation d'ingérence et de désinformation, sans pouvoir intervenir dans la réponse ou la contre-attaque a apporter, nous sommes loin de Taïwan qui répond à une désinformation en 2 heures et 200 mots, j'espère que l'impulsion donnée par la revue nationale stratégique sera de nature à rendre plus efficaces nos actions de contre-ingérence la passivité est une erreur qui nous a coûté très cher, je parle de l'opération de désinformation, dont l'armée française a été victime dans l'affaire de Bounty au Mali, en janvier, les leçons en ont été tirées, l'efficace riposte pour déjouer le stratagème de Wagner du charnier de Gossi l'a démontré, il nous faut maintenant assumer une posture plus offensive, y compris dans le domaine de la cybersécurité, il nous faut un nouvel ordre de bataille car les menaces de cybersécurité croissent, suivant un rythme exponentiel, l'augmentation des moyens humains et budgétaires du SGDSN cette année, comme les précédentes, doit être salué, mais malgré cela, la progression des attaques contre les services publics, les collectivités territoriales et les établissements de santé n'a pas été ralenti nos capacités techniques, notamment l'expertise de l'Annecy sont reconnus par nos partenaires, mais allons-nous nous contenter de regarder chaque année, le compteur s'affoler et tendre l'autre joue lorsque les hackeurs auront pas réalisé un hôpital de plus d'principaux partenaires américains et britanniques ont compris qu'allait entraver les cybercriminels sur leur terrain, c'est aussi prévenir les attaques avant qu'elles n'arrivent est ainsi prête pratiquer une forme de dissuasion numérique je formule donc la proposition que nous nous dotions d'une stratégie offensive face au cyber attaques que nous nous dotions d'un directeur national de la cybersécurité et que nous coordonnons avec nos principaux partenaires. Car c'est un combat sans frontières pour conclure, je voudrais insister sur 2 points : la nécessité de continuer à former tous les acteurs de la cybersécurité, à commencer par les simples utilisateurs et en conséquence rechercher les responsabilités des gestionnaires de collectivité ou d'administration s'ils n'ont pas suivi les recommandations en matière de sécurité informatique, à l'image de la sécurité incendie alerter sur la nocivité du paiement des rançons, ceux qui sont contraints de payer pour sauver leur entreprise doivent savoir qu'ils contribuent également au financement du terrorisme mer génère un avis favorable à l'adoption de ce volet des crédits merci merci. La parole est à monsieur Mickaël, rapporteur pour avis de la commission des Affaires étrangères pour 3 minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, sur les rapporteurs, chers collègues, mon collègue Olivier Cadic vient de vous exposer les aspects macro-de ce sujet cyber défense telle qu'il est traité dans le programme 129 je vais me concentrer pour ma part, sur la menace du quotidien envers les citoyens, les entreprises et les collectivités, si nous faisons de la plateforme si ma vie en ce point gouv un baromètre, nous constatons qu'elle a enregistré 2 millions et demi de visiteurs en 2021 soit 101 % de plus en un an que les grandes menaces demeure l'hameçonnage le piratage de comptes et le rançongiciel ça, ça ne change pas mais ce qui évolue d'une année l'autre, ce sont nos points de vigilance et nous tenons ici, a insisté sur 2 points saillants la nécessité absolue de faire monter en gamme, la sécurité informatique et la résilience dans les systèmes de santé d'une part et à prendre conscience des faiblesses identifiées dans les outre-mer, d'autre part, en effet, lorsque le système informatique de l'hôpital de Corbeny de l'hôpital, pardon de Corbeil-Essonnes se trouve paralysé par une attaque au rançongiciel, le véritable préjudice n'est pas le coup d'une rançon de 10 millions d'euros qu'un établissement hospitalier public et d'ailleurs dans l'incapacité de payer le vrai préjudice est bien plus large et peut remettre en cause notre sécurité nationale car la paralysie de tout un hôpital, c'est la nécessité de rediriger les patients vers d'autres établissements, avec le risque de perte de chance thérapeutique que cela implique et ce risque devient majeurs dans les outre-mer, imaginez une neutralisation du centre hospitalier dans une collectivité d'outre-mer, sans possibilité de redéploiement délit à proximité, par conséquent, nous alertons sur la nécessité de pérenniser et améliorer les nouveaux outils mis en oeuvre par le plan France relance tout d'abord la fin du plan France relance pose la question de la pérennité des Centres de réponse à incendie régionaux et sectoriels dit c'est Syrte à cet égard, il faut signaler que 12 régions métropolitaines sur 13 se sont inscrites dans le programme, à l'exception de la région Auvergne-Rhône-Alpes ensuite, se pose la question de la montée en puissance des centres de réponse sectorielles, d'abord pour les Outre-mer, nous l'avons évoqué et en métropole vers la sécurisation et la labellisation des moyens informatiques du secteur de la santé des collectivités territoriales et de l'industrie, il s'agit de mission prioritaire pour lesquels les moyens du plan de relance non encore engagées mais aussi les crédits dégagés pour 2023 doivent être fléché, enfin, il est proposé que la plateforme numérique Silbert malveillance Point gouv se transforme en un véritable sans véritable centre d'appels apte à traiter les incidents de 1er niveau et à rediriger les cas les plus graves à des prestataires locaux ou à Lancy quand il y a le feu, on appelle le dix-huit, par réflexe bien partager le S10 dispose de la compétence en matière de traitement des appels, celle-ci pourrait être expertisé en coordination évidemment avec l'si le GIP Acyma et les régions qui ont mis en place des Centres de réponse pour résumer, nous approuvons l'augmentation des moyens dans ce programme, non sans pointer les urgences que nous avons identifiés et les failles à combler, j'aimais comme mon collègue, un avis favorable à l'adoption de ce volet des crédits de la mission Direction de l'action du gouvernement, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est maintenant aux questeurs, Jean-Pierre Sueur, rapporteur pour avis de la commission des lois pour 3 minutes. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, présenté 35 pages et 6 budget en 3 minutes, n'a pas de sens, je le dis, chaque année, je le répète, s'agissant de la présidence de la République, je tiens également à informer le Sénat que monsieur le directeur de cabinet du président de la République a pour la 3ème année consécutive, refusé de recevoir personnellement votre rapporteur pour avis, pour des raisons que j'ignore s'agissant de la présidence de la République, les crédits augmentent de 4 9 % mais surtout les dépenses de fonctionnement augmentent de 18 millions, ce qui fait 12 61 %, soit nettement plus que l'inflation, il y a des dépenses très justifié ce sont celles qui relèvent de la sécurité du président de la République, sur lesquels les augmentations proposées nous paraissent tout à fait pertinente en revanche pour le reste, il y a beaucoup de flou, je cite le rapport qui nous a été envoyé par la présidence de la République, dit qu'il s'agit, je cite, d'un recalibrage réaliste devenu indispensable permettant de faire face aux coûts de gestion courante donc le recalibrage réalise devenu indispensable permettant de faire face, je ne vais pas tout relire mais c'est abscons, c'est de la langue de bois, quoi, donc, on est toujours dans l'incertitude par rapport à cette augmentation de dépenses de fonctionnement s'agissant du Conseil constitutionnel, naturellement, les dépenses se baisse et c'est très bien, mais c'est parce qu'il y aura ni présidentielles, les législatives, enfin en principe l'année prochaine pour ce qui est des QPC je salue l'initiative du Conseil constitutionnel qui a établi une base de données, on a plus de 1000 QPC dont Question prioritaire de constitutionnalité qui ont été étudiés par le Conseil, et d'autre part, j'ai cru devoir rappeler le vote du Sénat, par 322 voix sur 348 membres du Sénat selon lequel l'année dernière, nous avons décidé que il fallait que les ordonnances soient ratifiées par le Parlement de manière expresse et nous avons tenu à rappeler ceux-là à la sagesse du Conseil constitutionnel, enfin, monsieur le président, pour ce qui est de la Cour de justice de la République, il n'y a pas beaucoup de choses à dire, sinon que, il y a eu en un an 20119 recours présenté par rapport au Covid, je dis bien 20119 98 % d'entre eux proviennent d'un seul avocat qui a diffusé une plainte près rédigée sur Internet, ce qui a conduit à cette procédure, qui d'ailleurs a intéressé l'Ordre des avocats qui pose incontestablement problème moyennant quoi, la commission des lois vous propose de voter ces crédits. La parole est maintenant à monsieur Guy Bénard Roche, rapporteur pour avis de la commission des lois pour 3 minutes. C'est le président, monsieur le Ministre, chers collègues, la commission des lois et saisie pour avis des programmes soit 65 Conseil d'État et autres juridictions administratives et 164 Cour des comptes et autres juridictions financières de la mission Conseil contrôle de l'État, ces 2 programmes présentent des crédits inscrits au projet de loi de finances pour 2023 d'augmentation de leurs de 9 % et un schéma d'emplois également en hausse avec 41 équivalents temps plein pour les juridictions administratives et 5 équivalents temps plein pour la Cour des comptes, les juridictions administratives ont été confrontés en 2021, une forte reprise de l'augmentation des affaires reçu leur niveau dans les tribunaux administratifs a dépassé de près de 4 5 % celui déjà exceptionnellement élevé de l'année 2019 parallèlement les affaires en instance de plus de 2 ans en progressé dans les 2 niveaux de juridiction et le stock des dossiers en première instance a augmenté de 5 dans ces conditions, la programmation pluriannuelle qui prévoit la création de près de 200 emplois au bénéfice des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel d'ici 2027 et bienvenue, elle ne doit toutefois pas masquer les importantes difficultés de gestion qui s'annonce, en raison de la réforme de la haute fonction publique, en particulier des obligations de mobilité renforcée qui s'imposera désormais aux magistrats administratifs, par ailleurs, la commission des lois a estimé qu'une attention particulière devait être portée à l'organisation et au fonctionnement des services chargés de rendre les ordonnances de tri ou pour les cours administratives d'appel celle rejetant les requêtes manifestement dépourvu de fondement, compte tenu des volumes de dossiers qu'ils traitent et des conséquences d'une telle orientation pour le justiciable en 2021 ces ordonnances en moyenne 20 % des sorties devant des TA et 38 % devant les cours administratives d'appel, or les services chargés de les ordonnances repense souvent sur des assistants de justice et des vacataires, la décision qui sont formés en peu de temps, et fréquemment renouvelée, compte tenu de leur statut, de ce fait, il ne semble pas satisfaisant de se remettre au seul contrôle juridictionnel du Conseil d'État en cas de pourvoi, compte tenu du fait que certains justiciables peuvent y renoncer en raison de la nécessité de prendre un avocat au Conseil une supervision dédié par un magistrat expérimenté semble nécessaire, le métier d'agent de greffe a fortement évolué aussi au cours des dernières années, il recouvre de nombreuses fonctions et mal connu, et de nombreux postes ne sont pas pourvus par mobilité mais par un recours accru aux agents contractuels ou vacataires de longue durée, il est donc important de donner en 2023 des suites concrètes au rapport du groupe de travail sur l'avenir des grèves. S'agissant des juridictions financières, l'absence de Goya il y a eu bah supplémentaires alloués aux chambres régionales et territoriales des comptes, c'est d'être des inquiétudes quant à la capacité à assumer leur rôle en matière de contrôles de régularité des côtes et de lutte contre les enquêtes à la probité au niveau local et à nourrir par des desserrer la chauffe de contentieux de la Cour des comptes, le périmètre des compétences de ces juridictions s'est étendu de manière importante au cours des dernières années et le nord désorganise soumis à leur contrôle s'est multiplié en 2023 viendront également s'ajouter les nouvelles missions d'évaluation des politiques publiques territoriales, par ailleurs, le régime de responsabilité étant désormais répressif et de visant que les fautes de gestion les plus graves, il devra reposer sur des contrôles plus minutieux et de Bordeaux, des compétences techniques, plus il existe donc et d'inquiétude quant à la Bavière dans les chambres pour continuer à assumer leur rôle en matière de contrôles de régularité et de lutte contre les atteintes à la probité au niveau local, le projet de loi de finances pour 2023, c'est en fait évoluer les indicateurs de performance du programme j'aborderai cette question tout à l'heure lors de la présentation de l'amendement que j'ai déposé au nom de la commission des lois, en conclusion, monsieur le président,

C'est le président, Monsieur le Ministre, mes, mes chers collègues. Sur la mission Direction de l'action du gouvernement de programmes principaux : le programme 129 qui représente 86 % des crédits de de la mission et notre et notre rapporteur spécial a indiqué petite croissance mais largement justifiée par le contexte à la fois sécuritaire mais aussi technologique et le programme 308 qui est celui qui d'autre en crédit les, les, les autorités administratives indépendantes et pour lesquels il faut à la fois accompagner l'augmentation des périmètres de leur mission et d'émissions qui parfois prennent plus d'ampleur contre une du fonctionnement de de l'administration, les nouveautés principales cette année pour le programme 129 c'est la mise en place du code secrétariat général à la planification écologique pour quinze TP là le besoin de croissance de la dièse pour évaluer et encadrer l'évolution de la haute fonction publique, compte tenu de la réforme de la haute fonction publique la nécessité de renforcer le Haut Conseil pour le climat et enfin pour le SGE, le besoin de mieux suivre les le suivi des des consommations de crédits européens de faire du reporting dans le cadre du plan de relance pour avoir la meilleure capacité d'absorption possible des fonds européens, là où j'émettrai une réserve, c'est sûr, les ETP qui sont consacrés au CNR, dont nous savons ce que nous en pensons ici et au commissariat au Plan sur les questions de sécurité cybersécurité qui a largement été développé la lutte contre les fausses informations le nouveau cadre légal de renseignements qui exige aussi un certain nombre de moyens complémentaires pour logique et pour Losique enfin la question de 18 qui a été aussi évoquée par nos rapporteurs, il est bien effectivement d'identifier l'effet que News et les actes inamicaux, il serait mieux de pouvoir les entraver et de pouvoir avoir des réponses adéquates beaucoup d'évolution au cours des dernières des derniers temps en matière de de périmètre la fusion CSA Hadopi avec l'Arcom comme qui démarre, le défenseur des droits, qui a besoin de moyens complémentaires pour faire face, en particulier au déficit de fonctionnement d'administration d'accès au droit de dématérialisation, avec le besoin de moyens nouveaux pour former et accompagner les des délégués territoriaux, la CNIL, qui est absolument essentiel, là encore pour notre adaptation qui a fait face à un gros une grosse tension dans le domaine des, des, je note aussi qu'elle 25 millions d'euros de budget mais 214 millions de sanctions qui vont dans le budget de l'État puisque la CNIL arrive à sanctionner la CGLPL qui a aussi un un fonctionnement absolument nécessaire, en particulier dans la lutte pour identifier les les questions de dignité en termes de rétention et la CNCTR qui doit faire face à la mise en place de son nouveau cadre légal avec des moyens complémentaires, c'est la raison pour laquelle notre commission vous propose d'adopter les crédits de cette mission. Comment si chers collègue vu leur monsieur le Ministre, mes chers collègues, je vous propose que nous attaquions la DG en écoutant la présidente associée Nathalie Goulet je suspendrai après Nathalie Goulet. Pas d'opposition, je le vois, vous êtes tous contents allez madame la présidente, ça si c'est à vous pour quatre minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je souhaiterais m'attarder au sein de la mission, pouvoirs publics sur les dépenses de la présidence de la République qui me paraissent de nature à légitimer les démontre que les demandes que nous formulons pour nos concitoyens et les collectivités territoriales, l'inflation de l'année 2023 est estimé dans ce budget à 4,2 % les crédits de la présidence de la République au Mans augmente plus vite à 81 la dotation de la présidence sera donc en augmentation de 5,5 millions d'euros quand dans le même temps, les dotations des collectivités plafonne à une augmentation 2 fois inférieur, une augmentation en trompe-l oeil, un trompe l'oeil les dépenses élyséennes augmente de 3,9 % soit plus rapidement que les 3 5 accordées aux fonctionnaires du pays quant aux dépenses de fonctionnement pour lesquels les collectivités territoriales se voit imposer régime sec au travers du retour par une voix déguisée des contrats de Cahors avec des reprises financière à la clé la présidence augmente les siennes de 12,61 % à juste titre, le rapporteur général souligne la traduction budgétaire de l'augmentation des départs général les fluides énergétiques, les denrées alimentaires, les matériaux de rénovation plus surprenant est de constater que cette envolée de dépenses de fonctionnement et marqué par l'évolution des outils informatiques, singulièrement des opérations de maintenance préventive plus nombreuses et plus autre plus coûteuse, ces dépenses, nous les dénonçons non non dans leur nature et j'insiste sur ce point car nous partageons bien évidemment, la nécessaire lutte par exemple contre la cyber Crime criminalité mais nous les dénonçons dans leurs conditions de réalisation et l'augmentation du recours aux contractuels et à des entreprises extérieures pour assurer des missions régulières au sein de ces des institutions, ce recours accru ne doit pas être motivée par des raisons strictement budgétaires mais doit au contraire relevé uniquement de la stricte nécessité un plan de performance est prévue pour nous rassurer et concernent notamment les dépenses de déplacement pour un coût de 7 millions d'euros l'année précédente, un journal notait à juste titre que l'usage des engins de l'escadron de transport, d'entraînement et de calibration n'est plus notifié dans les documents budgétaires sûrement pour économiser quelques lignes de papier, gage de la sobriété de l'exécutif qu'il s'applique sans détour qu'il applique sans détour aux citoyennes et citoyens du pays, il est plus qu'indispensable que les services de l'État au 1er rang du duquel la présidence s'adapte à la demande des citoyens et des élus, à plus de transparence et concrétiser une ambition d'exemplarité, un mot tout de même sur le budget alloué au Conseil constitutionnel qui lui aussi est en baisse cette année, nous avons, je dois dire du mal à comprendre pour quelle raison les dépenses de fonctionnement sont cette année en diminution de près d'un tiers de millions cette année, contre 3 6 en n'a-t-il plus de n'a-t-il pas de locaux à chauffer ou d'agents à nourrir la situation du Conseil est intéressante car elle illustre un phénomène commun à l'ensemble des juridictions les dossiers augmente, mais les moyens humains ne suivent pas ou peu en progression constante depuis plusieurs années, les questions prioritaires de constitutionnalité sont un signe de démocratisation du droit constitutionnel, l'initiative de 2021 prévoyant de déployer un système d'information de la question prioritaire de constitutionnalité l'initiative du Conseil constitutionnel est louable car il permettra une meilleure information des citoyens en ce qui concerne les décisions prises par l'institution donc face à un budget, je dirais, en demi-teinte qui privilégie iniquité entre les crédits alloués à la présidence et le sort réservé à l'administration centrale du pays aux autres échelons de la puissance publique et surtout à nos concitoyennes et concitoyens, nous ne pouvons que nous abstenir sur cette mission. Merci madame la présidente, la parole est maintenant à madame Nathalie Goulet pour le groupe Union centriste pour six minutes. Monsieur le Ministre, si c'est les rapporteurs mes, mes chers collègues, moi aussi je vais vous parler de cyber criminalité, on ne compte plus les cyber attaques, on en a parlé beaucoup ce matin la filière cyber a été renforcée par l'augmentation du nombre de gendarmes et policiers une cyber patrouilleurs, ce qui est quand même une une bonne chose, Tracfin. Ah aussi développé une cellule notamment dédié à la délinquance financière est liée au au crypto-. Motif : le 23 novembre dernier, le Parlement européen subit une attaque informatique avec l'adoption d'un texte concernant la Russie, doyen Badinter les notes. Table vieillissant, parlent de leur affaire et de leur vie, dans leurs discours, moi, je voudrais vous parler de l'article du Sunday Time et des attaques et du piratage de mes comptes et de ma boîte GMail par le Qatar, ce qui n'était pas très agréable, je n'ai pas reçu à ce jour, un appel du service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères je ne sais pas non plus si la boîte du Sénat a été piraté, ce qui est quand même assez désagréable, j'espère que la justice fera évidemment toute la lumière sur cette affaire mais je voudrais revenir aussi en matière de cybercriminalité sur les problèmes liés aux cryptoactifs Monsieur le Ministre, parce que le ministre de l'Économie et des Finances a souhaité faire de la France une plateforme pour les cyber actif, je ne sais pas si la faillite de la plateforme FTX a ralenti ses élans mais je pense que en ce qui concerne cette question il faudra vraiment forcer sur la formation des cadres et des dirigeants sur cette ce question spécifique des cryptoactifs, sur laquelle j'ai le sentiment que ni les. Ni les autres ne sommes vraiment préparé, je crois qu'il faut faire de la cybercriminalité, une grande cause nationale Monsieur le Ministre, l'agence de l'Union européenne pour la cyber, c'est que la cyber sécurité a rendu le 23 novembre dernier un rapport sur les investissements des entreprises essentiel, essentiel, c'est-à-dire celles qui pourrait impacter l'économie et les prestataires numérique et la société de matières générales, ces entreprises ont dépensé 4 millions en 2021 contre 10 millions d'euros en 2020 pour leur protection, il y a là un problème et je crois que toutes ces questions sont sont liés, car un investissement moindre dans des mesures de notre rapporteur souligne enfin la nécessité pour le SG PR que je me suis fait prendre à mon propre piège doit faire prendre melon, le rapporteur, dit un solide discernement dans le recours aux cabinets privés, a fortiori sur un sujet aussi sensible que la transition et ne. je trouve cet avis intéressant, il prend en cause évidemment le travail excellentissime de notre commission d'enquête sur les cabinets privés et j'espère que pour aider ce secrétariat général à faire preuve de discernement le gouvernement, comme il s'y est engagé, fera mettre à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, la proposition de loi sur les cabinets privés qui a été voté au Sénat, les comités Théodule, on en voit encore beaucoup, dont on ne doute pas du tout qu'ils vont magnifier l'action publique, le Haut Conseil pour le climat, le secrétariat général à l'applique à la planification écologique tout ça fait preuve d'un manque de cohérence et probablement de coordination en tous les cas, il y a des doutes dans le cas du travail du du rapporteur, il faudra évidemment juger sur la durée, le travail de la délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'État la dièse créé il y a juste un an, par décret du 24 décembre 2021 chargé du vivier des cadres dirigeants supérieurs de l'État, alors là j'ai quand même une interrogation de ce ministre, comment, comment Rendez-vous compatible ce travail avec le fait de casser la haute fonction publique notamment diplomatiques avec la disparition un lundi de Pâques, du corps diplomatique et des grands corps de l'État, il faut quand même savoir ce qu'on veut, vous ne pouvez pas à la fois former des viviers et casser les outils, moi j'y vois quand même une incohérence, sauf à y placer les recalés du suffrage universel. enfin, que penser. De l'augmentation des Budgets consacrés à la participation citoyenne, cette participation citoyenne, sinon qu'au bout d'un moment, elle finit quand même par détourner les vrais sujets du Parlement, que ce soit le Conseil national de la refondation de la reconstruction et de tout ce que vous voulez des participations citoyenne, tout ça est un moyen supplémentaire de procrastiner et de détourner les sujets de la décision des parlementaires, je pense que ce n'est pas une mode, méthode de travail, encore une fois, ces sujets sont des sujets importants, nous allons néanmoins voté les Budgets de cette mission, monsieur le Ministre, j'attire votre attention sur les questions de cybercriminalité, comme l'ont fait mes collègues mais surtout sur plus de cohérence en ce qui concerne la formation et le respect qu'on doit à la haute fonction publique dans ce pays et notamment nos nos diplomates avec la fin du corps diplomatique, il me semble être une erreur absolument fondamental, je vous remercie. Merci, cher collègue, je vais su. Fendre la séance, elle sera reprise à 14 heures 30 pour la suite de l'examen d'émission, pouvoirs publics, Conseil et contrôle de l'État et direction de l'action du gouvernement, la séance est suspendue.